qui nous permet d'éviter tout risque d'une société de surveillance. Ensuite, et par exception, en raisonnant cas d'usage par cas d'usage, celui de garantir la sécurité des grands événements au cours desquels le risque terroriste est avéré. De fait, les multiples facettes des technologies biométriques soulèvent de nombreux enjeux éthiques en matière de liberté, de sécurité et de souveraineté. Parmi ces techniques, la reconnaissance faciale vise à reconnaître une personne sur la base des données de son visage. Les cas d'usage sont potentiellement illimités. Les deux premières entreprises mondiales spécialistes de cette technique sont françaises et leurs algorithmes sont désormais fiables à plus de 99 %.

comme des données « sensibles » au sens du RGPD, les données biométriques font l'objet d'une interdiction de traitement, lequel ne peut être mis en oeuvre que par exception, dans des cas très particuliers : avec le consentement exprès des personnes, pour protéger leurs intérêts vitaux ou sur la base d'un intérêt public important, comme le prévoit la directive relative à

Comme en matière de bioéthique, il s'agit de fixer dans la loi de grands interdits applicables à tous, en particulier aux acteurs publics : interdiction de la notation sociale ; interdiction de la catégorisation d'individus en fonction de l'origine ethnique, du sexe ou de l'orientation sexuelle, sauf dans le cadre de la recherche scientifique

La proposition de loi que nous vous présentons, traduisant en cela parfaitement l'esprit et la lettre du rapport d'information, prévoit qu'une fois les lignes rouges définies et garanties, certains cas d'usage exceptionnels peuvent légitimement être expérimentés- j'y insiste -dans le cadre d'un régime de contrôle extrêmement renforcé. D'où la proposition d'une loi d'expérimentation

L'expérimentation pourrait être autorisée pour trois ans, ce qui obligerait le Gouvernement et le Parlement à réévaluer le besoin et à recadrer éventuellement le dispositif en fonction des résultats obtenus, voire à le supprimer totalement. Afin que cette phase d'expérimentation soit utile serait mise en place, outre le contrôle parlementaire, une évaluation publique, conduite par un comité composé de scientifiques et de spécialistes de l'éthique indépendants dont les rapports seraient bien évidemment rendus publics.

de la reconnaissance biométrique, dans le cadre de consultations pour avis s'agissant des analyses d'impact et de contrôles du bon usage des dispositifs et des éventuels détournements de finalité.

permettre de manière subsidiaire, et uniquement pour la recherche d'auteurs ou de victimes potentielles des infractions les plus graves, l'exploitation d'images se rapportant à un périmètre spatio-temporel limité, sous le contrôle du magistrat chargé de l'enquête ou de l'instruction. En deuxième lieu, pour instituer une nouvelle technique de renseignement afin que les services du premier cercle puissent traiter les images issues de la voie publique à l'aide de systèmes de reconnaissance, uniquement à des fins de protection de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, de défense nationale et de prévention du terrorisme. En troisième lieu, pour créer un cadre juridique permettant, de manière subsidiaire et par exception, le recours ciblé et limité dans le temps à des systèmes de reconnaissance biométrique sur la voie publique en temps réel- c'est ce point qui fait débat -sur la base d'une menace préalablement identifiée, vue de la sécurisation des grands événements face à un risque terroriste ou d'atteinte grave à la sécurité des personnes. De nombreuses garanties entourent ce dispositif, qu'il s'agisse de la formation spécifique des agents utilisateurs ou de l'encadrement des modalités de développement et de déploiement du dispositif : nombre limité de caméras dédiées, distinctes de celles des systèmes de vidéoprotection, ce qui permet de circonscrire fortement le périmètre géographique et temporel.

en répartissant différemment les dispositions du texte, afin de créer un bloc précisant les garanties apportées et les interdits posés. Il a également souhaité interdire l'identification à distance sans consentement : avec le texte modifié, l'utilisation de la reconnaissance faciale devrait être exclusivement prévue par des dispositions législatives, et non réglementaires.

Succédant à ce socle très important de garanties, un autre bloc définit le régime de contrôle et d'autorisation, le rôle du Parlement, qui doit être central, et les usages possibles de ces technologies.

à l'unanimité. Je souligne ce consensus parce que l'extrême sensibilité de la question traitée ne garantissait pas à l'avance un tel résultat. Si les recommandations de nos collègues se sont ainsi imposées à nous, c'est grâce au discernement, à la prudence, aux interrogations, aux scrupules et même aux doutes qui les ont inspirés. Avec eux, notre ambition est simple : protéger efficacement la vie privée des Français et garantir leurs libertés, sans pour autant renoncer totalement aux possibilités ouvertes par l'intelligence artificielle dans le traitement de données biométriques pour sauver des vies menacées par le terrorisme ou la grande criminalité. la voie était étroite, mais nos collègues ont su l'explorer avec sagesse ; dès lors, votre commission des lois n'avait plus qu'à l'emprunter et à la prolonger pour renforcer encore les garanties imaginées dans leur proposition de loi, en précisant les interdits posés, puis en resserrant le cadre juridique imaginé pour la mise en oeuvre d'exceptions fortement restreintes et drastiquement contrôlées. De quoi s'agit-il ? De l'utilisation d'une technologie permettant de reconnaître une personne photographiée ou filmée dans l'espace public au travers de la mise en équations numériques de son visage et le rapprochement des données ainsi obtenues avec les données déjà détenues sur la même personne. Il est ainsi possible de savoir si une personne se prévaut d'une fausse identité ou si une personne est présente parmi d'autres individus dans un lieu public donné. Et l'on peut procéder soit dans l'instant pour une action de prévention ou de poursuite immédiate, soit dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une opération de renseignement. Le parti susceptible d'être tiré de cette technologie est immense, comme sont immenses les risques qu'elle comporte du fait de son caractère extraordinairement intrusif. Tombée entre les mains de la police d'un régime dictatorial, elle peut devenir l'instrument d'un contrôle social généralisé. Utilisée à titre exceptionnel et de manière restrictive dans un régime démocratique respectueux de l'État de droit, elle peut ponctuellement présenter un intérêt réel pour la protection des citoyens, à condition que les principes et les règles encadrant son utilisation soient à la hauteur des libertés que nous, législateurs, en particulier le Sénat de la République, devons absolument faire prévaloir. J'ai abordé ces questions avec à l'esprit quelques références communément partagées : nous savons bien que la marche de la science conduit depuis toujours à des découvertes ambivalentes, le meilleur côtoyant le pire. De la maîtrise du feu jusqu'à celle de l'atome, nous avons constamment été confrontés à ces interrogations auxquelles nul n'a jamais mieux répondu que Rabelais, avec qui nous disons désormais que « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Mes chers collègues, c'est à nous d'apporter la conscience nécessaire à la maîtrise et au contrôle des usages de l'intelligence artificielle, aujourd'hui pour la reconnaissance faciale biométrique. L'Union européenne travaille sur le même sujet. Un règlement européen est en gestation. Il s'inspire de principes largement communs aux nôtres, ce qui n'est pas surprenant, car la France conserve une place déterminante dans le processus législatif européen. Il pourrait aboutir en 2025. Nous vous proposons de ne pas attendre cette échéance pour agir. La France, comme elle l'a fait avec Bernard Kouchner et Simone Veil voilà trente ans dans un autre domaine où science et éthique se confrontaient- la bioéthique -, peut et donc doit être précurseur. C'est en effet pour nous une vocation sans cesse renouvelée que d'affirmer des principes fondamentaux en matière de libertés, dont d'autres pourront ensuite s'inspirer. Et cela nous mettra en position de force dans la négociation européenne en cours. Nous avons bien évidemment tenu compte du travail accompli à Bruxelles et à Strasbourg et des réflexions engagées par la Cnil dès 2019, ainsi que des conclusions de nombreux rapports, le plus récent, très riche, étant celui de nos collègues députés Philippe Gosselin- de la Manche ! -et Philippe Latombe. Nous pensons maintenant être en mesure d'engager un processus législatif fécond, susceptible d'aboutir à l'Assemblée nationale. Les principes que nous vous proposons d'adopter sont relativement simples. Il y a d'abord un principe absolu, très clair, qui ne peut donc souffrir aucune exception : il s'agit de l'interdiction de toute exploitation d'images issues de la vidéosurveillance dans le cadre d'un contrôle social à la chinoise, avec classement des individus en fonction de leur comportement dans l'espace public en vue de les avantager ou, au contraire, de les pénaliser. Il y a ensuite des principes auxquels seul le législateur pourra déroger, dans des conditions strictement limitées et contrôlées interdiction de la reconnaissance faciale en temps réel à distance sans consentement, par exemple dans le cadre de la vidéosurveillance ; interdiction aussi de l'exploitation par reconnaissance faciale d'images déjà détenues par la justice ou la police, sauf exception qui serait alors décidée par la loi et non par décret, comme dans certains cas aujourd'hui. Ces principes étant établis, le texte prévoit ensuite les possibilités de dérogations, ainsi que les finalités et le régime de celles-ci. Les dérogations devront être prévues directement par le Parlement. Elles seront expérimentales, d'une durée de trois ans, placées sous le contrôle du Parlement, obéissant aux principes de proportionnalité, de nécessité et de subsidiarité, et devront utiliser des logiciels de traitement configurés sous la responsabilité de l'État et individuellement autorisés,

La Cnil, justement, comme l'ont proposé Philippe Gosselin et Philippe Latombe, sera consacrée comme autorité régulatrice des usages de l'intelligence artificielle. Sa composition sera complétée pour associer les autorités de régulation de l'audiovisuel et des télécommunications à ses missions. Le contrôle d'accès par la reconnaissance faciale pourra être utilisé lors de grands événements, comme nous souhaitons le faire pour les jeux Olympiques mais de manière limitée à certaines catégories d'intervenants professionnels ou bénévoles, à certains lieux, avec une information préalable des intéressés, sans possibilité d'intégrer les riverains à ces modalités d'accès s'ils n'ont pas donné leur consentement, et seulement en cas de menace particulièrement grave pour la sécurité. La reconnaissance faciale pourra être aussi utilisée pour le besoin d'enquêtes judiciaires. D'abord, par la validation législative de la possibilité d'utiliser la reconnaissance biométrique pour identifier des personnes inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires. Ensuite, pour l'exploitation d'images de vidéosurveillance déjà recueillies, et cela en vue de réprimer le terrorisme, les trafics d'armes et les atteintes aux personnes punies de plus de cinq années d'emprisonnement, ainsi que pour la recherche de criminels en fuite ou de personnes disparues. Par ailleurs, dans des conditions tout à fait exceptionnelles, limitées aux crimes les plus graves, à la disparition de mineurs, à la lutte contre le terrorisme et à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, la justice pourra recueillir des images grâce à des caméras dédiées et les exploiter en temps réel la reconnaissance faciale en vue d'assurer le succès de l'enquête, au lieu de devoir utiliser seulement des images préexistantes. il faudra l'autorisation d'un magistrat, qui ne pourra être renouvelée au-delà de quarante-huit heures qu'avec l'accord du juge des libertés et de la détention. Seuls des officiers de police judiciaire, qui plus est spécialement habilités, pourront mettre en oeuvre le traitement. Enfin, l'utilisation de la reconnaissance faciale dans des activités de police administrative, c'est-à-dire de police préventive, préventive, sous l'autorité du Gouvernement, se fera, sur ma proposition, dans des conditions centralisées et non sur simple décision du préfet. Il reviendra au Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et sous le contrôle du Conseil d'État, de prendre la décision- c'est le système robuste de la loi de 2015 relative au Mes chers collègues, les questions que nous avons à traiter aujourd'hui sont en apparence techniques et juridiques ; pourtant elles sont plus encore d'essence politique et éthique. L'approche de la commission des lois conforte, je le crois, les intentions équilibrées des auteurs de ce texte, tout en étendant les garanties qu'ils y avaient déjà inscrites. Le caractère expérimental de la proposition de loi, comme nous l'avions déjà décidé en matière de terrorisme, présente l'intérêt de suivre l'évolution d'une technologie que l'on dit mature, mais qui n'est pas à l'abri d'erreurs. Il nous permettra aussi d'évaluer les éventuelles difficultés de mise en oeuvre, de nous appuyer sur une jurisprudence et, finalement, de vérifier que nous avons trouvé le bon équilibre. Puisque nous avons l'audace de cette première étape, ayons aussi l'humilité d'accepter que notre oeuvre ne soit pas pleinement aboutie et de prévoir qu'elle puisse être encore améliorée à la lumière de l'expérience.

La sensibilité de ce sujet nous impose donc prudence et mesure dans les évolutions que nous pouvons opérer. Vous savez combien le Gouvernement est déterminé à faire avancer vite les sujets qui l'exigent, comme la transformation écologique ou la formation des jeunes, en passant par la souveraineté énergétique. Mais il est des sujets dont la complexité justifie peut-être que nous différions quelque peu les décisions définitives, même lorsque l'on pense disposer de propositions judicieuses. La reconnaissance biométrique en fait partie. Je rappelle que vous venez de voter le cadre juridique de l'expérimentation du recours à l'intelligence artificielle (IA) pour concourir à la sécurisation des jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Dans ce cadre, le Gouvernement et le Sénat ont fait preuve de prudence et de mesure. Le Gouvernement, d'abord, qui a proposé un texte extrêmement encadré, avec des garanties nombreuses, une durée très limitée, des finalités de recours à l'IA réduites et l'exclusion de la reconnaissance faciale.

Certes, un important travail transpartisan avait été mené sous la férule des sénateurs Marc-Philippe Daubresse, Arnaud de Belenet et Jérôme Durain, dont je salue l'implication et la hauteur de vue.

En effet, il nous semble important de nous interroger sur la temporalité de cette proposition de loi d'un point de vue politique, juridique et opérationnel. D'un point de vue politique, d'abord. Légiférer maintenant sur la reconnaissance biométrique, précisément alors que va s'engager la négociation entre le Conseil et le Parlement européen sur le projet de règlement sur l'intelligence artificielle (RIA), dont le périmètre est encore assez mouvant, risquerait d'affaiblir notre position de négociation. En effet, il pourrait exister un décalage inévitable entre nos positions à Bruxelles et le texte voté à Paris. Du point de vue de la cohérence et de la lisibilité de notre droit, ensuite. ensuite. Cette concomitance de calendriers nous obligera en tout état de cause à revenir sur une législation nationale à peine votée, le règlement devant être adopté à l'échelon européen d'ici à la fin de l'année et traduit en en droit interne en 2025 au plus tard. Cette configuration est loin d'être optimale en termes de prévisibilité de la norme, pour une expérimentation dont la durée est fixée à trois ans, vous en conviendrez. Je sais Je sais combien votre assemblée a été sensible à la nécessité d'offrir à nos acteurs industriels un cadre juridique stabilisé et clair, permettant à la France de disposer de solutions souveraines.

D'un point de vue opérationnel, enfin. Le tempo de la proposition ne nous paraît en effet pas le plus opportun. Toutes nos forces sont mobilisées vers la sécurisation des jeux Olympiques Depuis que vous avez donné mandat au Gouvernement pour expérimenter l'IA, le ministère de l'intérieur travaille jour et nuit, d'ailleurs en très bonne intelligence avec la Cnil, afin d'être au rendez-vous de cette expérimentation. Celle-ci est complexe et soulève des questions opérationnelles importantes avec des défis de coordination entre tous les acteurs de la sécurité des futurs grands événements- État, communes, RATP, SNCF. Il ne paraît ni opportun ni possible de distraire les forces de sécurité de ce chantier majeur pour s'investir dans la reconnaissance faciale, dont je rappelle que le Gouvernement n'avait, de son propre chef, pas proposé l'utilisation à l'occasion des L'expérimentation proposée dans ce texte serait nécessairement décevante : sur les trois années dont il disposerait, le Gouvernement n'aurait en réalité ni le temps ni les ressources pour s'y engager pleinement. D'autant qu'il aurait un peu le même raisonnement que les entreprises nationales dans ce domaine : entre un RIA en fin de négociation, appelé à devenir rapidement la référence européenne, et un cadre français dont l'extinction est prévue à court terme, les deux ne disant pas exactement la même chose, le bon sens commandera de faire plutôt application des règles européennes. En outre, en cette matière, le recours à la biométrie à des fins de police administrative et judiciaire ne peut se prendre de manière isolée en ce qu'il s'inscrit dans une stratégie plus large de politique de sécurité. La biométrie ne constitue qu'une brique devant s'intégrer dans une doctrine opérationnelle et dans un cadre juridique d'action des forces de sécurité intérieure. Je crois que les auditions que vous avez menées,

il est difficile, voire impossible, de se prononcer dans l'absolu sur le recours à la biométrie sans avoir une vision claire de toute la chaîne stratégique et de l'ensemble du cadre technique. s'il est en théorie intéressant d'appliquer la reconnaissance faciale des caméras pour vérifier si un individu dangereux se trouve dans un lieu où il n'est pas censé être, cela soulève en pratique des questions extrêmement lourdes. Les réponses à y apporter doivent conditionner la conception de la norme et non l'inverse non l'inverse : qui décide de la liste des gens dangereux ? Quelles caméras dans un contexte où les communes et les acteurs privés disposent de 98 % du parc dans notre pays ? Quels services peuvent mettre en oeuvre cette technologie ? Un cadre juridique qui serait trop en décalage avec la « vraie vie » des services de sécurité et d'enquête risque de rater sa cible, car les possibilités qu'il offrira ne répondront pas À cet égard, si je salue le travail du rapporteur, il me semble que l'État est le mieux à même de déterminer les éléments de doctrine opérationnelle, ce qui permettrait en outre de bénéficier du regard du Conseil d'État et de la Cnil. De façon générale, les auteurs de la proposition de loi partent du présupposé que les usages de la biométrie dans l'espace public soulèvent tous les mêmes questions, alors que les problématiques opérationnelles et les besoins de légiférer ne nous semblent pas correspondre. Ainsi, nous regrettons que les auteurs ne distinguent pas plus nettement l'usage le plus complexe, à savoir la reconnaissance faciale en temps réel à des fins de police administrative, d'autres usages beaucoup moins attentatoires comme la recherche d'un individu dans le cadre d'une enquête. Ce faisant, votre commission a voulu que relève de la loi tout traitement recourant à la biométrie, ce qui rigidifiera considérablement le droit des traitements de données. Cette idée est à rebours des exigences européennes dans ce domaine, qui nous font de plus en plus obligation de recueillir et d'inscrire de la donnée biométrique pour assurer l'interopérabilité et la fiabilisation des fichiers. De plus, cette approche est frontalement contraire à la recommandation n° 18 de votre rapport d'information, qui visait à « mettre en place, par la prise de décrets en Conseil d'État, la possibilité pour les forces de sécurité nationale d'interroger à l'occasion d'une enquête judiciaire ou dans un cadre de renseignement certains fichiers de police par le biais d'éléments biométriques ». Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, si le Gouvernement salue la volonté de votre assemblée de traiter ces sujets- je salue particulièrement le sénateur Daubresse, dont nous connaissons l'engagement sur les sujets régaliens et de sécurité et son souci de garantir au ministère de l'intérieur les moyens de son action action -et partage l'utilité de les traiter, nous ne sommes pas pleinement convaincus de l'opportunité de légiférer maintenant. Il paraîtrait plus pertinent au ministre de l'intérieur et à moi-même de renvoyer à un projet de loi

Houlala ! C'est souvent la réaction que suscite l'évocation de la reconnaissance biométrique et d'un débat sur le sujet. Est-ce en

que certaines initiatives gouvernementales prennent la forme de propositions de loi. Souvent ! Il arrive encore que certaines propositions de loi soient amendées et améliorées par le Gouvernement dans le cadre d'un échange avec le Parlement. J'espère que c'est ce que nous sommes en train de commencer à faire.

proposition de loi tend à transcrire les conclusions des travaux de la mission d'information précitée et vise à ce titre deux objectifs principaux répondre aux besoins de régulation de ce système de surveillance, d'autre part, permettre aux pouvoirs publics d'utiliser à titre exceptionnel ces technologies, de les comprendre, de les maîtriser, d'en tester l'utilité. Le principe est l'interdiction, l'expérimentation l'exception. Remanié par la commission des lois, l'article 1 tend à poser clairement l'interdit du traitement des données biométriques aux fins d'identifier une personne à distance dans l'espace public et dans les espaces accessibles au public,

elles, sont très encadrées : limitées à trois ans, elles sont régulièrement évaluées et dans le cadre d'un rapport public et par le Parlement. Elles sont soumises à un régime de contrôle : les usages de la reconnaissance biométrique dans l'espace public répondent à une procédure d'autorisation spécifique, de la part des magistrats pour les usages judiciaires et de celle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour les usages administratifs. concerne les usages judiciaires, la commission a estimé que le recours à la reconnaissance biométrique ne devait être expérimenté que dans le cadre des enquêtes et des instructions portant sur des infractions d'une exceptionnelle gravité.

que les cas extrêmes : enquêtes portant sur des faits de terrorisme ou d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, sur des infractions relatives à la criminalité organisée ou sur des disparitions de personnes mineures. la commission a entendu renforcer au maximum le régime de contrôle de cette expérimentation ainsi que les garanties associées. Elle a ainsi soumis l'usage à une autorisation expresse de l'autorité judiciaire qui devra préciser préciser l'origine et la nature des données exploitées. Elle a également confié au seul juge des libertés et de la détention le soin de procéder au renouvellement de l'autorisation de recourir aux traitements biométriques en question. Pour ce qui est des usages administratifs, la commission a restreint le champ de l'expérimentation en prévoyant que le système d'authentification biométrique obligatoire ne pourrait concerner les habitants des zones concernées. Elle a aussi précisé que seul l'État pourrait mettre en oeuvre les traitements de données biométriques utilisés dans le cadre de cette expérimentation. C'est important à souligner, car il s'agit bien bien de notre souveraineté : il ne faudrait pas que toute une série de technologies, faute de législation dédiée, partent à l'étranger. Il faut plus précisément que l'État maîtrise lesdites technologies pour pouvoir exercer son contrôle légitime et protéger nos libertés publiques.

grâce aux initiatives de notre rapporteur, a réussi à aller plus loin. J'y vois là un gage considérable donné à ceux qui pourraient s'inquiéter pour nos libertés. J'y vois

mon « sentiment profond que le fait de présenter l'innovation technologique comme une solution évidente demeure une chimère potentiellement dangereuse ». Et voilà que vous proposez dans ce nouveau texte d'expérimenter le recours à la biométrie.

en fonction de leur comportement. Ce dispositif repose sur une collecte de données des personnes sur leur comportement dans la rue ou dans les transports. Tout cela donne une note qui permet d'identifier la qualité du citoyen et d'en déduire le périmètre de ses droits. Pour y parvenir, l'usage de la biométrie est essentiel Nous sommes déjà dans ce que les scénarios d'anticipation les plus préoccupants pouvaient proposer voilà à peine quelques années. Aussi, j'aime à répéter à cette tribune combien le groupe RDSE est fermement attaché aux libertés. À cet égard, les limites fixées tant par les auteurs de la proposition de loi que par notre rapporteur sont évidemment à saluer, d'autant qu'il est inenvisageable de ne pas les inscrire dans la loi. Elles tiennent compte des inquiétudes et des risques encourus par notre société. Je pense à l'interdiction de catégoriser des personnes sur la base de leurs données biométriques, à l'interdiction de noter des personnes, toujours sur la base de ces données, ou encore à l'interdiction des systèmes de reconnaissance biométrique en temps réel ou dans l'espace public. Seulement, tout le monde sait bien que le législateur peut défaire ce qu'il a fait. Ces garde-fous sont certes indispensables, mais ils seront insuffisants le jour où il sera question de les faire sauter. J'en viens maintenant à la série d'expérimentations que proposent les auteurs du texte. Chacun s'accordera autour de la nécessité de sécuriser les événements particulièrement exposés à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes. Je pense bien évidemment aux jeux Olympiques et Paralympiques. Chacun s'accordera également à vouloir faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces mêmes infractions et la recherche de leurs auteurs. En quelques mots, les expérimentations proposées visent toutes des buts légitimes dont la gravité justifie certaines innovations en matière de surveillance ou d'investigation. Si ces dispositifs devaient être institués, il faudrait en effet les accompagner, comme le proposent les auteurs du texte, d'un comité scientifique et éthique chargé d'évaluer régulièrement l'application des mesures.

Aussi, malgré des réserves assez importantes quant au développement de la biométrie, et même si la position de notre groupe n'est pas unanime- c'est souvent le cas -, une partie majoritaire d'entre nous votera en faveur de cette

et une première traduction législative d'un encadrement de son utilisation qui manquait cruellement à notre arsenal juridique. Ce texte une réelle ambition : celle de garantir le juste équilibre entre outils technologiques de sécurité collective et respect de l'État de droit et des libertés fondamentales, dans l'intérêt de nos concitoyens. loi viennent poser un principe d'interdiction qui fera l'objet d'une liste d'exceptions strictement encadrées par des procédures et des garanties de surveillance collectives et transparentes. Ce texte est le résultat d'une réflexion parlementaire qui a fait l'objet de trois rapports ces dernières années. son travail remarquable, notre rapporteur, le questeur Philippe Bas, est venu renforcer et parfaire l'esprit de cette initiative législative. Le Sénat a ainsi l'occasion de faire entrer la France dans le nouveau millénaire en matière de sécurité.

Après les vaccins qui inoculeraient des puces brevetées par Bill Gates, la vidéoprotection avec reconnaissance faciale dans l'espace public violerait notre intimité C'est une possibilité, d'où un encadrement strict de son utilisation. Pourtant, avouons-le, il y a là un paradoxe insensé : nous acceptons chaque jour de céder à des multinationales étrangères la moindre donnée personnelle récoltée au travers de nos téléphones, de nos téléviseurs et de nos enceintes connectées, ou encore, désormais, de nos voitures intelligentes, mais nous refusons que l'État régalien assure notre sécurité par tout moyen technologique, comme la vidéoprotection avec reconnaissance faciale, alors même que telle est sa mission.

Mes chers collègues, la reconnaissance faciale et biométrique n'est qu'une goutte d'eau et un balbutiement dans les avancées de l'intelligence artificielle. Nous voilà rassurés

Permettez-moi d'être très inquiet quand je constate le sous-équipement des principales grandes villes françaises en matière de vidéoprotection. Pourtant, c'est dans ces métropoles que se concentrent la criminalité, la violence et le terrorisme.

pour Toulouse. Dans le même temps, deux capitales européennes majeures, Londres et Berlin, en dénombrent respectivement 180 et 110, toujours pour 10 000 habitants. Nous sommes clairement en retard par rapport à nos voisins. Comment imaginer que Paris et Marseille, qui accueilleront dans les prochains mois la Coupe du monde de rugby, une messe du pape ou encore les jeux Olympiques, soient quasiment nues en matière de vidéoprotection ? Au-delà de ces grands événements, rappelons tout de même que la France est le pays le plus touristique du monde avec 89 millions de visiteurs par an. La gare du Nord est la plus fréquentée d'Europe avec 700 000 voyageurs quotidiens. Nous devons garantir une protection dans l'espace public à la mesure de notre attractivité. La France doit s'adapter à son époque : on ne peut lutter contre les délinquants et contre les terroristes du XXI siècle avec les outils désuets et obsolètes du milieu du XXsiècle. Pour conclure, je citerai Clemenceau, qui fit tant pour notre sécurité collective : « Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. » La parole

Cet outil permet d'identifier un individu grâce à un panel de caractéristiques qui lui sont propres. L'intelligence artificielle connaît un essor fulgurant. Notre rôle de législateur prend tout son sens dans ce domaine où tout va très vite. Nous avons besoin d'un droit solide et protecteur qui saura s'adapter aux évolutions C'est indispensable pour protéger nos droits fondamentaux et nos libertés individuelles. Dans notre pays, la reconnaissance biométrique est très limitée et le droit n'est pas du tout adapté.

La reconnaissance biométrique est là, elle existe ; elle peut être utile pour améliorer la sécurité dans l'espace public et lors de grands événements. Dès lors, pourquoi s'en priver ? Développons intelligemment ce nouvel outil, faisons-le de manière sécurisée, avec un modèle qui nous convient. Fixons nous-mêmes les règles et les limites que nous souhaitons nous imposer.

cela a été souligné, ce débat représente également un enjeu de gestion des données. Google, Facebook, TikTok : ces plateformes américaines ou chinoises captent à longueur de journée des données relatives à nos populations. Nous peinons à voir émerger des outils européens en la matière. Ne prenons pas le même retard sur la reconnaissance biométrique Nous saluons la Commission européenne, qui s'est saisie de la question de l'intelligence artificielle avec l'. Je rejoins l'avis du rapporteur : nous ne pouvons attendre 2025 et l'entrée en vigueur de ce futur règlement européen. Tout va très vite : beaucoup de nos voisins ont déjà recours à la reconnaissance biométrique. Nous ne sommes pas les États-Unis, où la pratique est encadrée de manière plutôt vague ; nous ne sommes certainement pas non plus la Chine, ... Pas encore ! ... où des millions de caméras intelligentes sévissent chaque jour et notent les individus.

L'expérimentation sur une durée de trois ans va dans le bon sens. Nous devons évaluer ces mécanismes avant une potentielle pérennisation. La subsidiarité introduite dans les mécanismes est gage de préservation des libertés. La limitation des expérimentations à des cas très précis, à caractère exceptionnel, est centrale. Ces mécanismes sont cruciaux dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et dans la défense des intérêts de la Nation. L'expérimentation prévue concernant les grands événements sportifs et ses conditions de mise en oeuvre sont des pistes de réflexion intéressantes pour l'avenir. Trouver l'équilibre entre la sécurité des Français et le respect de leurs libertés est la ligne de crête sur laquelle nous devons en permanence avancer.

créer un cadre juridique expérimental permettant, par exception et de manière strictement subsidiaire, le recours ciblé et limité dans le temps à des systèmes de reconnaissance biométrique sur la voie publique,

n'allait pas assez loin dans les innovations en matière de surveillance. Notons les précautions, les circonlocutions et les périphrases : elles ne sont pas anodines et résument en réalité les faux-semblants qui sous-tendent le présent texte. En vérité, En vérité, le procédé est toujours le même lorsqu'il s'agit de technologies de fichage et de surveillance de masse : à la prudence initiale se substituent la généralisation et la fin des garde-fous. la fin des garde-fous. Les prélèvements ADN, par exemple, ont été introduits dans notre droit en 1998 à la suite de l'affaire Guy Georges et concernaient à l'époque uniquement les condamnés définitifs pour agression sexuelle. Vingt-cinq ans plus tard, le fichier national automatisé des empreintes génétiques répertorie 3 millions d'individus, avec une écrasante majorité de personnes non condamnées. Nous ne comptons plus les prises d'empreintes génétiques pour des participations à des manifestations, par exemple ; refuser de s'y soumettre constitue désormais un délit, passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Ficher l'ADN des militants politiques est devenu coutumier ! La vidéosurveillance a connu le même essor au travers d'un usage exponentiel, qui en a rendu la pratique massive.

que l'on nous jure strictement encadrées, pour aboutir invariablement à des généralisations. Nos libertés publiques deviennent secondaires pour les apprentis sorciers de la société de surveillance.

sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste ait dénoncé l'utilisation du terrorisme comme justification politique pour adopter des technologies à haut risque. Qu'importe que la Défenseure des droits souligne un « risque inhérent d'atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données ». Qu'importe que le (MIT) révèle que les technologies de surveillance automatisées présentent des préjugés liés au sexe et à la couleur de peau. Il nous faudrait innover dans la société de contrôle, toujours plus loin, toujours plus fort, sans jamais réfléchir au modèle de société que cela induit. Que contient ce texte ? Une forte dose d'hypocrisie. En effet, son article poser un cadre très strict d'interdictions pour empêcher la catégorisation, la notation ou la reconnaissance des personnes par les technologies de biométrie, le tout assorti d'un contrôle sérieux du Parlement, de la Cnil ou de la CNCTR. On aurait pu s'arrêter là, avec quelques sanctions pour des usages illégaux. Pourtant, que contient le reste du texte ? Une liste d'exceptions à cette interdiction générale. La biométrie ? Jamais, sauf pour contrôler l'accès aux grands événements, pour permettre l'exploitation d'images afin de retrouver des auteurs ou des victimes d'infractions, pour surveiller des foules en direct lors d'événements dits à risque ou ou encore pour aider aux investigations des services de renseignement dans la lutte contre le terrorisme. La liste est déjà longue, mais elle sera trop courte pour un prochain gouvernement qui pourra introduire à souhait des exceptions supplémentaires. À partir du moment où vous acceptez, avec ce texte, la dissémination, la prolifération de ces technologies, vous devrez assumer un usage qui deviendra général, n'en doutez pas. Ce texte est un cadeau de bienvenue à un prochain gouvernement plus autoritaire qui n'aura qu'à pérenniser l'usage de la biométrie en rallongeant la liste des usages possibles. Celles et ceux qui sont attachés à la devise républicaine, notamment au premier terme gravé au fronton de nos mairies, celui de « liberté », devraient être horrifiés par ce texte. Les garde-fous n'y changeront rien : l'autorisation, même partielle, de ces technologies ne fera qu'en multiplier le développement et l'usage. La société de surveillance mettra à mal notre démocratie. L'usage politique de ces technologies ne sera pas entravé par les garde-fous. Les dérives politiques de la surveillance policière sont déjà très concrètes. La se faisait encore l'écho la semaine dernière d'un bras de fer entre Matignon et Beauvau quant à la surveillance et la mise sur écoute de militants écologistes. L'enjeu n'est pas seulement sécuritaire, il est aussi économique. Beaucoup appellent- de telles ambitions ont été énoncées très clairement durant les débats sur la loi d'orientation soutenir et développer des champions français de la technosécurité. Au nom de la défense des libertés publiques, nous refusons le projet de société que vous défendez avec ce texte : une société du fichage, du flicage, de l'abolition du privé de l'intime ; un continuum de sécurité, qui considère tout comme une donnée à traiter, jusqu'au phénotype même des individus ; un carcan indépassable, qui n'a qu'une visée, le contrôle, partout et tout le temps. C'est pourquoi nous vous proposerons la suppression de la plupart des articles de cette

portant sur la reconnaissance biométrique dans l'espace public. Issu des propositions formulées par une mission d'information de la commission des lois, ce texte vise, d'une part, à fixer des lignes rouges pour faire obstacle à une société de surveillance, d'autre part, à expérimenter de nouveaux cas d'usage de cette technologie, qui croît exponentiellement grâce aux algorithmes d'apprentissage. Nous le savons, l'opinion publique est polarisée entre ceux qui craignent l'usage poussé des technologies biométriques en raison de leur nature attentatoire aux libertés et ceux qui soulignent davantage ses bénéfices potentiels pour la sécurité de tous. La reconnaissance biométrique dans l'espace public n'est effectivement pas un dispositif anodin. Elle fait partie de ces outils qui relèvent d'un choix de société et qui requièrent donc une attention et une évaluation toutes particulières. En effet, ses applications possibles sont illimitées : elles peuvent dépasser le seul prisme sécuritaire pour rythmer un simple acte de la vie courante ou une activité commerciale. Dès lors, permettre l'usage de telles technologies sans instaurer de garde-fous est dangereux. Des exemples au-delà de nos frontières nous montrent comment cet usage comporte une part de risque, notamment lorsqu'il est utilisé par un régime totalitaire contre ses propres citoyens. Nous avons tous en tête l'exemple de la Chine, où la reconnaissance faciale rythme le moindre acte de la vie quotidienne - obtenir une ligne de téléphone portable, faciliter l'enregistrement dans un hôtel, identifier des élèves qui sèchent les cours

À cet égard, l'analyse des services de la Cnil, qui a été présentée à la commission des lois par son secrétaire général, Louis Dutheillet de Lamothe, est aussi éclairante qu'alarmante. Selon ce dernier, alors que l'expérimentation des technologies biométriques ne devrait être réalisée qu'« avec une extrême prudence et de manière progressive », la proposition de loi que nous examinons élargit de manière considérable et d'un seul coup les cas d'usage ». Comme il le rappelle, choisir d'expérimenter, c'est déjà choisir de créer. Contrairement aux recommandations des services de la Cnil, la commission des lois a fait le choix de maintenir les dispositions relatives à la reconnaissance biométrique en temps réel, ce que regrettons vivement. Selon M. Dutheillet de Lamothe, l'identification en temps réel dans l'espace public à titre expérimental marquerait « une rupture fondamentale pour l'exercice de nos libertés publiques, alors que nous n'avons pas encore de recul sur l'efficacité et l'utilité de la biométrie dans les autres cas cas d'usage ». Et je n'évoque pas les risques avérés d'erreurs d'identification, les biais discriminatoires, le risque d'inhibition dans l'exercice des droits ou libertés fondamentales ou encore le risque de sécurité informatique. Par conséquent, avant d'étudier la possibilité de recourir à cette technologie, nous estimons préférable de prendre le temps de tester l'emploi des caméras augmentées, sans reconnaissance faciale, dont l'expérimentation est prévue par l'article 10 de la très récente loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. convient donc de faire le bilan de cette expérimentation qui se déroulera au cours des jeux Olympiques et Paralympiques, à partir du 26 juillet 2024, avant d'aller plus loin quant au développement de la reconnaissance faciale.

et je m'inclus dans ce « nous », à débattre des mesures concernant la vidéoprotection algorithmique lors des jeux Olympiques et à répéter, souvent avec sincérité : « non, il n'y aura pas de reconnaissance faciale aux JO ». Cela était dit avec sincérité pour plusieurs raisons : nous étions nombreux à penser qu'il était trop tôt, que les critiques exprimées dans la société à l'égard de l'utilisation des algorithmes sans données biométriques créaient suffisamment de réticences et qu'il convenait d'éviter d'aller encore plus loin avec la reconnaissance faciale. De manière plus pragmatique, de nombreux acteurs nous disent qu'il est trop tard, que mettre en place les systèmes de reconnaissance faciale prend du temps et que rien ne serait de toute façon opérationnel pour les JO. Je pense que ces messages, que nous avons nous-mêmes répétés, ont été entendus. Permettez-moi d'en rappeler quelques-uns. « Nous nous félicitons de ce que la ligne rouge de la reconnaissance faciale n'ait pas été franchie dans le projet de loi déposé par le Gouvernement », déclarait la rapporteure de la commission des lois sur le récent projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques. « Je suis opposé à la reconnaissance faciale », affirmait Gérald Darmanin, auditionné par notre commission. Nous ne voulons pas de la reconnaissance faciale ni de l'utilisation de données et de systèmes d'identification biométrique pour ces Jeux. Non seulement ces procédés ne nous semblent pas nécessaires sur le plan opérationnel, mais, surtout, les autres dispositifs prévus permettront, à eux seuls, un saut qualitatif en matière de prévention et de lutte contre les troubles à l'ordre public », déclarait Amélie Oudéa-Castéra à l'Assemblée nationale. l'ai bien compris, certaines de ces citations sont soumises à interprétation, voire à une date limite de validité. Je comprends ces subtilités. Après tout, j'ai moi-même signé le rapport de la commission des lois sur la reconnaissance faciale, avant de refuser de signer la proposition de loi qui en découlait. Permettez-moi de vous expliquer mon raisonnement personnel avant de vous confier la position de mon groupe sur cette proposition de loi. Je ne crois pas que la reconnaissance faciale, telle qu'elle est perçue par les auteurs du texte, dont je connais les intentions, la qualité du travail et le souci de prendre de grandes comme par notre rapporteur, constitue un danger en soi. C'est une technologie qui commence à être efficace, même si elle conserve quelques faiblesses. Elle est déjà utilisée par nos citoyens pour certains de leurs actes quotidiens-

M. le rapporteur estime que cela interviendra trop tardivement. Je pense au contraire qu'il ne sert à rien de se précipiter sur un sujet éthique qui aura des conséquences sur plusieurs décennies. Je considère que ce sujet mériterait un débat national d'envergure, oserais-je dire une convention citoyenne ? Je ne crois pas que nos compatriotes soient par nature opposants ou partisans de cette technologie et je ne préjuge pas des conclusions qui pourraient en sortir. Je suis un fervent défenseur de la démocratie parlementaire, mais je crois que, sur certains sujets pour lesquels l'acceptabilité est essentielle, il importe de mettre en place des processus de décision associant le plus grand nombre possible

La réécriture opérée par M. Bas a ses vertus, la volonté d'encadrer cette technologie étant louable. Toutefois, nous pensons que l'heure n'est pas venue. Par ailleurs, en matière technologique, l'effet cliquet n'est jamais loin, précédente ayant évoqué l'audition du secrétaire général de la Cnil. Aujourd'hui, nous repoussons le modèle chinois de reconnaissance faciale, comme nous repoussions hier l'internet à la chinoise, protégé derrière son grand. Pourtant, de plus en plus de voix jalousent les possibilités offertes par l'internet chinois pour protéger les mineurs ou censurer des contenus dangereux. Sommes-nous certains, mes chers collègues, que le modèle chinois de reconnaissance faciale constituera toujours un repoussoir dans dix ans ?

Pour avoir débattu de l'utilité de cette technologie avec des dizaines de personnes ces dernières années, je retiens quelques limites qui nous permettront de relativiser l'urgence de notre débat. Premièrement, la reconnaissance faciale n'est pas une recette miracle. Oui, elle sera utile dans certains cas enlèvements de personnes, menace terroriste identifiée - j'insiste sur le terme « identifiée » -, recherche de personnes dangereuses précises. Elle ne fera pas disparaître l'ensemble des menaces. Certes, elle sera utile dans la résolution d'enquêtes, mais il faut garder à l'esprit que la vidéoprotection elle-même n'a pas fait disparaître la criminalité dans notre pays. Même si elle est utile, elle a ses limites, et la Cour des comptes ne s'est pas privée de le rappeler à de multiples reprises. La vidéoprotection et la reconnaissance faciale ne vont pas sans intervention humaine. Dans des exemples dramatiques, encore très récents, ce sont bien des interventions humaines qui ont permis de mettre fin au drame qui se déroulait. Aucune caméra, avec ou sans reconnaissance faciale, n'aurait pu empêcher ce qui s'est passé. Un acteur du renseignement me disait, de façon un peu triviale, « ce n'est pas parce que j'identifie celui qui a rayé ma voiture sur le parking que ma voiture est réparée ». Il n'y aura

Face aux bouleversements de l'intelligence artificielle croisée avec les données biométriques, il nous semble prudent d'avancer conjointement avec l'Europe. Vous le comprendrez, et le regretterez peut-être, nous ne soutiendrons pas ce texte.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, si la pratique de la surveillance des populations par l'État est ancienne, sa massification, sa sophistication et sa banalisation interrogent. Fichage massif de nos concitoyens, des organisations syndicales, des syndicalistes et des militants, déploiement incontrôlé de la vidéosurveillance, qu'elle soit traditionnelle ou algorithmique, usage de drones, marquage des manifestants, activation à distance des téléphones portables dans un but de géolocalisation, mais aussi activation à distance de la caméra et du micro de ces mêmes téléphones, scanners corporels La panoplie des mesures de surveillance, sous couvert de justification sécuritaire, s'enrichit de manière inquiétante, pour ne pas dire glaçante, et ce dans l'apathie générale. Ce qui, hier, relevait de la dystopie se concrétise pas à pas, sous nos yeux, sans aucun débat public. Pire, sous couvert d'écarter le risque d'une société de surveillance, le texte dont nous débattons aujourd'hui tend à instaurer le principe d'une telle surveillance, en se cachant derrière l'impératif de « préserver nos intérêts économiques en développant des outils techniques français qui améliorent la sécurité sans nuire aux libertés ». Et les jeux Olympiques ou autres « méga-événements » sont autant de chevaux de Troie « pour faire progresser des politiques qu'il aurait été difficile, voire impossible, de mettre en place en temps normal », comme le rappellent très justement de nombreuses ONG. C'est ainsi que ce texte vise, sous couvert d'expérimentation, dans une logique de prévention des risques, de lutte contre des menaces, supposées ou avérées, ou d'efficacité des enquêtes, de banaliser la vidéosurveillance automatisée. Cette surveillance massive de l'espace public a pour objet de détecter des comportements prétendument anormaux, l'identification par reconnaissance faciale en temps réel. Comme pour d'autres systèmes de surveillance par le passé, tout en reconnaissant le caractère intrusif des technologies biométriques, l'argument avancé pour les mettre est place est l'impossibilité « de se priver de la reconnaissance faciale dans des cas particulièrement graves, afin de garantir la sécurité de nos concitoyens, à condition que son déploiement, exceptionnel, soit entouré des garanties nécessaires ». pas « nous attarder sur les dangers réels de cette technologie en matière d'atteinte à la vie privée, sur les risques de développement d'une société de surveillance à la chinoise ou encore sur les erreurs possibles d'identification. présente des avantages dont il serait dommage de se priver définitivement. Elle permet notamment de prévenir des attentats ou encore de retrouver des criminels. » Notons-le, cette technologie est aussi la source de juteux revenus pour de nombreux acteurs privés. Nous parlons d'un marché en pleine expansion, qui pèsera près de 76 milliards de dollars dans le monde à l'horizon 2025. c'est au contraire des risques que font courir ces technologies et de la société que nous voulons qu'il faut débattre avant toute chose. Nous savons que ces dispositifs comportent des risques de discrimination, d'erreur, d'atteinte aux libertés fondamentales que nous ne pouvons balayer d'un revers de la C'est ce que nous confirme la Cnil, en pointant le fait que « les bases de données utilisées pour le calibrage des algorithmes - les femmes, les gens de couleur, les personnes différentes - sont moins bien identifiées par les intelligences artificielles, faisant peser le risque de leur occasionner plus de contrôles, moins de libertés. De plus, comme le souligne La Quadrature du Net, « les comportements dits " suspects " ne sont que la matérialisation de choix politiques, subjectifs et discriminatoires, qui se focalisent sur les personnes passant le plus de temps dans la rue. Qu'elle soit humaine ou algorithmique, l'interprétation des images est toujours dictée par des critères sociaux et moraux, et l'ajout d'une couche logicielle n'y change rien. » Enfin, ne nous y trompons pas, ces dix dernières années, toutes les mesures d'exception expérimentales ont fini, d'une manière ou d'une autre, par entrer dans le droit commun et par s'étendre à l'ensemble de la population et à toutes les situations. Depuis près de vingt ans, avec une accélération certaine ces dernières années, nous sommes enfermés dans des politiques sécuritaires dont l'efficacité n'a pas été prouvée. Les outils de surveillance se renforcent

chaque repli de la vie, autorité indolore et invisible et pourtant confusément acceptée. » Ne laissons pas l'exigence de sécurité briser le rêve de liberté

mais également servir la politique de répression d'un régime totalitaire. Son usage fait la une de l'actualité à quelques mois de la Coupe du monde de rugby en septembre prochain et des jeux Olympiques et Paralympiques Ne faut-il pas avoir peur de cette technologie potentiellement redoutable ? Rappelez-vous, le 16 avril dernier, la République islamique d'Iran a annoncé la mise en place d'une politique répressive pour lutter contre le non-port du voile. Pour arriver Pour arriver à ses fins, le régime des mollahs a annoncé l'introduction du système de reconnaissance faciale pour traquer ces femmes, militantes de la liberté. En Chine populaire, dans un pays qui maîtrise parfaitement cette technologie, la reconnaissance faciale a été généralisée au point que les autorités sont en mesure d'identifier dans la rue chaque individu, de connaître le solde de son compte bancaire, de procéder à la filature et à l'arrestation de celui ou de celle n'ayant pas payé son reliquat d'impôts

C'est dans ce contexte que, lors de l'examen au Sénat, en janvier dernier, du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques de Paris, la question de la reconnaissance biométrique s'est posée à la représentation nationale. En effet, 2024 sera une année où la France accueillera des sportifs et supporters du monde entier. Il serait terrible pour notre image que la menace terroriste ou la criminalité organisée viennent ternir cette période. Cela nous a permis de prendre conscience du vide juridique existant en droit français sur ce sujet. Il était donc urgent de légiférer et cette proposition de loi vient donner un cadre légal à l'usage de cette pratique. Pour cela, je remercie vivement mes collègues Marc-Philippe Daubresse, Arnaud de Belenet et Bruno Retailleau de nous présenter aujourd'hui ce texte. Un rapport d'information publié le 30 mars 2023 par quatre sénateurs de la commission des affaires européennes du Sénat a pour autant qualifié de « pratique à haut risque » la mise en place de la reconnaissance biométrique dans l'espace public, invitant le législateur à l'interdire totalement, sauf raison très exceptionnelle. Le texte qui vient aujourd'hui devant le Sénat tient compte de toutes ces préoccupations. Sur le fond, il précise, dès son article 1, que la reconnaissance biométrique est limitée par plusieurs lignes rouges. Il vise à interdire formellement la catégorisation, la notation et la reconnaissance biométrique des personnes physiques dans l'espace public. Je salue également le travail de la commission des lois et de son rapporteur Philippe Bas, qui a ajouté l'interdiction de l'identification dans l'espace public. Ces interdictions posent les bases d'une garantie de maintien des libertés, empêchant notre pays de sombrer dans une société de surveillance généralisée. Cela étant, il est nécessaire de se doter de tous les moyens que la technologie nous offre pour protéger les Français des attaques terroristes ou de la criminalité grandissante. il est proposé d'expérimenter pour trois ans un système de reconnaissance biométrique. Les différentes exceptions au principe d'interdiction seraient obligatoirement autorisées par la loi et l'application réglementaire se ferait après avis de la Commission nationale de de l'informatique et des libertés ou de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. En ce qui concerne l'utilisation d'images en temps réel, cette pratique serait limitée aux actions antiterroristes, afin d'éviter une attaque sur des civils innocents.

terroriste. L'utilisation d'images pour des enquêtes judiciaires, quant à elle, ne pourra se faire qu'après autorisation de l'autorité judiciaire afin de lutter contre la grande criminalité ou de rechercher des fugitifs ou des victimes d'enlèvement. Enfin, pour des événements particuliers ayant lieu sur la voie publique comme les jeux Olympiques, par exemple, ce système pourra être mis en place pour des actions de police administrative, donc préventive, lorsqu'une menace grave planera sur ledit événement. pas en détail tous les points de la proposition de loi, celle-ci arrive à point nommé. Elle me semble constituer un bon équilibre entre la nécessaire garantie des droits fondamentaux d'une démocratie comme la France et le défi d'une protection efficace de nos concitoyens. Ce texte, je l'espère, servira de base et d'exemple pour nos homologues européens en matière d'utilisation de la reconnaissance biométrique.

Le texte issu des travaux de la commission, qui sera soumis au vote du Sénat, exprime de façon très didactique la prise en compte des interrogations légitimes de certains élus sur les possibles dérives de la reconnaissance biométrique dans l'espace public et organise un dispositif légal garant de la sécurité des citoyens et des libertés publiques.

est à M. Thomas Dossus. Parce qu'elles ciblent le plus souvent les caractéristiques des individus qui les exposent à des discriminations, les technologies biométriques et la généralisation de leur usage sont susceptibles d'amplifier, pour certains groupes sociaux, les discriminations systémiques opérant au sein de la société. En d'autres termes, ces technologies sont biaisées. Lorsqu'elles sont déployées, elles ciblent en priorité les personnes pauvres, car la surveillance est basée sur des critères sociaux, en visant prioritairement les personnes se trouvant souvent dans la rue par manque de ressources. Outre les risques d'abus policiers, de tels biais contribuent aussi à engendrer un contrôle au faciès automatisé. Nous demandons donc d'interdire clairement la catégorisation et la notation d'individus sur la base de leur origine ethnique,

Ainsi, en janvier de cette année, un manifestant contre la réforme des retraites est passé en comparution pour avoir refusé de donner ses empreintes génétiques lors de son arrestation. Qui peut s'habituer à ce qu'on fiche l'ADN des militants politiques ou syndicaux ? Qu'est-ce qui nous garantit que la surveillance biométrique ne suivra pas ce même chemin ? Rien ! Certainement pas l'expérience que nous avons des évolutions législatives analogues ! C'est pourquoi nous souhaitons inscrire en toutes lettres dans la loi que la pérennisation ne va pas de soi et que le débat sur ces technologies a besoin de contradictoire.

Cet amendement vise à réintroduire dans la loi un principe de transparence relatif au développement des logiciels de traitement. En effet, il faut regretter que des garanties relatives à leur développement et à l'organisation du traitement des données biométriques, prévues dans la version initiale de cette proposition de loi, aient été supprimées au profit d'un simple renvoi à un décret en Conseil d'État. Pourtant, le législateur ne saurait consentir à cet abandon de compétence au profit du pouvoir réglementaire, par ailleurs susceptible de censure constitutionnelle. L'intervention du législateur est nécessaire dans ce domaine, car la reconnaissance biométrique résulte d'indissociables aspects immatériels et matériels. Cet abandon de compétence serait d'autant plus dommageable que des exigences européennes seront directement applicables sans que le législateur français se saisisse de ce sujet et fixe ses propres garanties. De manière concrète, enfin, il est nécessaire d'aider les autorités administratives compétentes dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle déontologique.

pendant une durée de quatre mois à compter de l'enregistrement des images. Il est par ailleurs prévu dans cet alinéa que ces images soient détruites au bout de trois ans après la promulgation de la loi. la promulgation de la loi. Les algorithmes, pour fonctionner correctement, ont besoin de données d'apprentissage. En l'espèce, pour la biométrie, ils ont besoin de voir et d'analyser des personnes afin de s'entraîner. Ce seront donc des personnes présentes dans l'espace public qui seront, sans leur consentement, des cobayes pour cet apprentissage. Ce n'est Ce n'est pas acceptable. Les libertés publiques n'ont pas à être un terrain d'entraînement ou d'expérimentation. Par ailleurs, le texte vise à prévoir que des entreprises privées puissent être chargées de développer des traitements biométriques. Cela signifie que leur activité et leurs revenus seraient donc assurés par des personnes non consentantes dans l'espace public. Même si des garde-fous sont érigés, même si la destruction des données est prévue, il y a là un glissement démocratique

au genre ou au type de couleur de peau. En analysant un logiciel de reconnaissance faciale, les chercheurs ont découvert un taux d'erreur de 0,8 % pour des hommes à la peau claire et de 34,7 % pour des femmes à la peau foncée. Par ailleurs, comme je l'ai déjà souligné, ce texte vise à prévoir que des entreprises privées puissent être chargées de développer des traitements biométriques. C'est une aubaine pour ces entreprises, puisque le marché de la vidéosurveillance automatisée au niveau mondial représentait, en 2020, plus de 11 milliards de dollars. Nous ne voulons certainement pas rendre ces technologies plus performantes et permettre aux entreprises de s'enrichir en exploitant la vie privée des personnes. C'est la raison pour laquelle nous proposons au contraire de remplacer le dispositif d'amélioration en trompe-l'oeil par un alinéa visant à indiquer que les critères sur lesquels se fondent ces traitements biométriques devront être disponibles en et que les données utilisées dans le cadre de ces traitements ne pourront être cédées ni vendues. parole est à M. Thomas Dossus. Comme je n'ai eu de cesse de le rappeler dans cet hémicycle, les technologies biométriques comportent des risques unanimement dénoncés par les autorités indépendantes, comme la Défenseure des droits ou la Cnil. Selon le rapport de 2021 de la Défenseure des droits sur les technologies biométriques, l'utilisation de la reconnaissance biométrique comporte un risque inhérent d'atteinte au droit et au respect de la vie privée, ainsi qu'à la protection des données. peut entraîner des discriminations, voire les amplifier. Pour la Cnil, la reconnaissance biométrique est particulièrement intrusive et comporte un certain nombre de risques pour la protection des données et de la vie privée. Face à ces risques indéniables dans la vie privée des personnes, nous proposons de renforcer les garanties pour les enregistrements utilisés à des fins pédagogiques en assurant l'anonymat des personnes figurant dans ces échantillons. Quel est l'avis de la commission ? L'amendement

par l'expérimentation, alors les risques d'erreurs qu'il s'agit justement d'éviter seront maintenus, au lieu d'être réduits. J'émets donc un avis défavorable.

prévoir que, avant d'utiliser les données issues de traitement biométrique par reconnaissance faciale pour des formations, il faudrait anonymiser les images recueillies. Mais notre texte interdit précisément d'utiliser ces données

des outils des forces de sécurité intérieure est incompatible avec l'exigence de sécurité. La confidentialité de leur fonctionnement technique est la condition de leur efficacité. À défaut, les délinquants et criminels s'en serviront à l'insu des forces de sécurité intérieure.

présenter l'amendement n° 6. L'article 2 tend à déroger, à titre expérimental, à l'interdiction de l'usage de l'authentification biométrique pour de grands événements, afin de permettre de contrôler l'accès aux zones. On arrive ici au coeur de la présente proposition de loi, au coeur de son hypocrisie,

L'expérimentation est une stratégie utilisée pour permettre un premier contact entre les pouvoirs publics et ces méthodes de surveillance biométriques. L'enjeu,, est d'ancrer ces technologies dans les territoires et de les normaliser dans notre environnement. Leur existence physique rapide des frontières extérieures (Parafe) dans les aéroports est un exemple de déploiement visant à banaliser ces technologies. C'est précisément l'objet de cet article 2, à savoir créer un phénomène d'accoutumance pour l'accès dans les stades ou les concerts. La pratique entrera ainsi plus facilement dans les moeurs. C'est ce que nous souhaitons éviter. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de cet article

ne pourront s'appliquer aux habitants des zones concernées par la mise en place de ce système. Ceux-ci devront donc disposer d'un moyen de substitution pour rejoindre leur domicile.

prévu que les riverains d'un grand événement ne seraient pas assujettis à cette expérimentation de la

qu'ils sont bien résidents de cette rue, on contrôlera alors leur identité, comme on le fait depuis toujours pour assurer la sécurité d'un lieu public en cas de menaces criminelles ou terroristes. En tout état de cause, après mûre délibération, la commission a émis Mme la ministre.

ou la victime d'une infraction sur les images recueillies dans le cadre d'investigations. Malgré les garanties supplémentaires ajoutées en commission, notre groupe s'oppose par principe à l'utilisation automatisée des données biométriques. Les garde-fous issus de la commission ne tiendront pas longtemps les antécédents de généralisation de ce genre de pratiques sont connus. Aujourd'hui, on met le doigt dans un engrenage sur lequel il sera difficile de revenir. Pour éviter l'effet de cliquet évoqué par mon collègue Durain, nous proposons donc la suppression de cet article.

Or ce fichier, dont nous avions d'ailleurs dénoncé la création, est tentaculaire : près de 19 millions de fiches sont présentes dans ce mégafichier, qui contient des informations à la fois sur les personnes mises en cause- peu importe qu'elles aient été condamnées ou non sur les témoins et sur les victimes impliquées dans les enquêtes. On se retrouve ainsi dans une situation où le recours à des logiciels d'analyse d'images automatisée serait rendu nécessaire, car le TAJ est devenu gigantesque, qu'il ne peut plus être exploité à son plein potentiel par des humains. Une surveillance de masse- le fichage généralisé -rend nécessaire une autre surveillance de masse- la reconnaissance faciale généralisée -, selon La Quadrature du Net. C'est la raison pour laquelle

crimes d'atteintes aux personnes punis de plus de cinq ans de prison, pour des agressions terroristes, pour la recherche de disparus, pour la recherche de criminels. Les conditions sont donc très

Nous avons pris des précautions qui n'existaient pas jusqu'à présent, puisque la consultation des antécédents judiciaires se fait sur la base d'un décret. Nous avons décidé qu'elle ne pourrait se faire que sur la base de la loi, mais encore faut-il le prévoir explicitement, et c'est ce que nous faisons. Nous sommes donc opposés à cet amendement.

La protection de nos concitoyens et des intérêts de la Nation est l'affaire de tous. En l'état, les réponses apportées par ce texte pour y parvenir font fi des erreurs et des biais des technologies biométriques, qui sont mal conçues peuvent entraîner l'aggravation des maux qu'elles prétendent combattre. Le développement expérimental de cette société de surveillance se fait au mépris des droits et des libertés collectives. Placée en garde-fou, la consultation pour avis de la Cnil ne constitue pas une garantie suffisante. En effet, en poussant la Cnil à accompagner les entreprises dans le développement de technologies biométriques, les auteurs de cette proposition de loi laissent à penser qu'une société de surveillance vertueuse est possible. Nous pensons exactement l'inverse : chaque pouce de terrain perdu pour nos libertés publiques nous rapproche des régimes

de la commission prévoit une décision du Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sous le contrôle du Conseil d'État. Les garanties sont donc maximales ! Par ailleurs, il s'agit uniquement de la lutte contre le terrorisme. Seuls les services chargés de la sécurité intérieure pourront mobiliser l'instrument de la reconnaissance faciale. C'est la raison pour laquelle la commission a considéré que ces amendements n'étaient plus justifiés, compte tenu de l'importance des garanties offertes, lesquelles reposent sur l'expérience acquise

de principe sur cet article, mais de lourdes réserves sur le dispositif envisagé. La technique de renseignement créée par cet article ne répond, à mon avis, à aucun besoin clairement défini. Soit l'objectif est de sécuriser un grand événement en empêchant l'accès aux individus suivis par les services de renseignement, et dans ce cas le recours à une technique de renseignement semble en pratique très compliqué. Soit l'objectif est de localiser en urgence un individu présentant une menace imminente pour l'ordre public, et, là encore, le dispositif ne paraît pas adapté. Il serait plus opportun d'autoriser l'exploitation des caméras de vidéoprotection, plutôt que de s'appuyer sur des caméras dédiées, dont le déploiement serait complexe dans une situation d'urgence et la couverture géographique probablement peu pertinente.

dans la discussion générale, il existe actuellement un conflit entre Beauvau et Matignon sur la notion de terrorisme. Matignon, pour l'instant, bloque les demandes

qui pourrait l'arrêter. Ce n'est pas notre modèle de société. Nos libertés publiques sont menacées par la dissémination et la prolifération de technologies de surveillance. Leur interdiction doit doit être un principe absolu. La reconnaissance biométrique, imparfaite, peut entraîner des erreurs de raisonnement aux conséquences multiples et potentiellement graves, telles que des arrestations erronées par les forces de l'ordre. En s'intéressant aux profils des personnes victimes de ces erreurs, la Défenseure des droits a bien insisté sur ces risques : il s'agissait majoritairement de personnes issues de groupes discriminés ou vulnérables, en raison des biais discriminatoires des algorithmes sur lesquels reposent ces technologies. J'insiste sur ce point : les enquêteurs ont suffisamment de moyens de surveillance à leur disposition pour ne pas avoir recours à un énième outil qui n'a pas fait ses preuves et qui comporte une grande marge d'erreur d'appréciation.

par une surveillance qui doit permettre d'identifier les auteurs d'un crime particulièrement grave. Je veux préciser que si cette possibilité d'emploi de la technologie de la reconnaissance faciale ne doit en aucun cas se généraliser, il nous paraît possible de l'expérimenter, à condition de le faire de manière extrêmement restrictive. C'est la raison pour laquelle les finalités de l'expérimentation ne pourront être que des enquêtes portant sur des actes de terrorisme, des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, des infractions relatives à la grande criminalité organisée et la disparition d'enfants qui auraient été enlevés. Bien sûr, si l'on veut prolonger au-delà de cette surveillance exercée sous le contrôle d'un juge, il faudra le demander à un juge des libertés et de la détention (JLD). Ce dernier vérifiera évidemment que l'enjeu est tel que se priver du recours à la reconnaissance faciale serait une perte de chance

du Gouvernement ? Faire de la reconnaissance faciale pour des finalités judiciaires répond en réalité à un vrai besoin. Pour autant, le dispositif envisagé ne nous paraît pas suffisamment opérationnel. La commission des lois a notamment supprimé la possibilité d'avoir recours à cette technologie afin d'identifier une personne en fuite, alors qu'il s'agit là de l'un des intérêts majeurs et suffisamment légitimes de ce dispositif.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous commençons cet après-midi l'examen de la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle. Permettez-moi tout d'abord de revenir sur le titre de cette proposition de loi. de cette proposition de loi. Oui, nous pensons que la réforme de l'audiovisuel public est une condition de la préservation de notre souveraineté audiovisuelle, dont chacun perçoit bien qu'elle est menacée, ou tout au moins questionnée. La réaffirmation de notre souveraineté audiovisuelle est également une condition de la préservation de notre audiovisuel public, qui réclame une profonde révision de la loi de 1986, pour que les nombreux verrous qui le pénalisent par rapport aux plateformes Nous pensons qu'il est urgent d'agir, non pas pour renforcer les contraintes sur les acteurs français, comme cela a souvent été le cas au cours des dernières années, mais, au contraire, pour libérer leur capacité à transformer leur modèle et à proposer des offres de programmes sur tous les supports. Le paysage a beaucoup changé depuis l'arrivée de Netflix en 2014. Les services de vidéo à la demande et les services proposant un accès illimité à la musique ont profondément modifié les usages de chacun d'entre nous. Il ne faut pas oublier certaines applications de partage de vidéos, comme YouTube et TikTok, qui sont devenues les univers préférentiels de la jeunesse. Selon des données qui nous ont été transmises au cours des auditions, il apparaît déjà que, en soirée, l'audience de ces sites de partage de vidéos est supérieure à l'audience de la télévision pour les jeunes. La télévision et la radio sont-elles condamnées à s'adresser aux générations les plus anciennes, donc, à terme, à disparaître ?

Mais le voulons-nous vraiment ? À quand remonte la dernière grande réforme audiovisuelle ? Alors même que les révolutions technologiques et d'usage s'enchaînent à un rythme inédit, nous sommes encore en train de nous interroger sur la réponse à apporter aux premières évolutions que, déjà, les suivantes arrivent. Ainsi, l'apparition des nouveaux acteurs et la numérisation de l'audiovisuel sont encore en train de produire leurs effets, en percutant notre modèle, que l'intelligence artificielle apparaît, suscitant de nouvelles questions et fragilisant encore nos organisations. Combien de temps faudra-t-il avant que les pouvoirs publics ne donnent un cap et n'apportent enfin les réponses aux attentes des acteurs du secteur, eux qui subissent de plein fouet ces évolutions ? Depuis une quinzaine d'années, plusieurs gouvernements ont annoncé la mise en chantier d'une grande réforme de la loi du 30 septembre 1986, mais tous ont renoncé devant l'obstacle, face aux pressions des groupes d'intérêts et aux corporatismes, mais aussi, il faut bien en convenir, faute d'avoir une vision claire du chemin à suivre. à suivre. Réformer la loi de 1986, ce n'est pas remettre en cause les principes fondamentaux de cette loi, auxquels nous sommes tous attachés. s'agit de permettre aux acteurs, publics comme privés, de faire face à de nouveaux concurrents, à la puissance financière incomparable et qui, pour de nombreux aspects, ne sont pas soumis à la législation française C'est tout le sens des propositions que je formule dans le chapitre II de ce texte, afin de lutter contre les asymétries de concurrence. Cette vision sur l'avenir de l'audiovisuel, en particulier public, nous y travaillons ici, au Sénat, depuis de nombreuses années. Dois-je rappeler les travaux de notre commission de la culture menés en partenariat avec la commission des finances en 2015, qui ont donné lieu au fameux rapport d'information de nos collègues Jean-Pierre Leleux et André Gattolin, puis au rapport d'information de nos collègues Jean-Raymond Hugonet et Roger Karoutchi, publié l'année dernière ? J'y insiste, ces rapports d'information portaient à chaque fois sur le financement des sociétés de l'audiovisuel public et concluaient qu'il était impossible de séparer le financement de l'organisation et de la gouvernance. Nous pensons toujours que ces trois aspects sont inséparables. Je n'oublie pas la dimension européenne de notre réflexion, qui s'est appuyée sur un colloque organisé en 2018 au Sénat, l'initiative de Catherine Morin-Desailly, avec la participation des présidents de la BBC, de la RAI, de la RTBF et de la RTS. Tous ces travaux nous ont convaincus qu'il était indispensable de donner plus de force à notre audiovisuel public, en regroupant ses talents dans une même structure, en confiant le soin de la piloter à une personnalité ayant une grande expérience des médias et en prévoyant des moyens suffisants dans la durée, afin de garantir son indépendance. Le rapport de nos collègues députés Jean-Jacques Gaultier et Quentin Bataillon n'aboutit pas à d'autres conclusions. Ils ont indiqué qu'ils étaient d'accord à 95 % avec notre proposition de loi. J'ajouterai que les 5 % qui manquent ne nous semblent pas des obstacles insurmontables. Comme la plupart de vos prédécesseurs, à l'exception de Franck Riester, vous avez choisi, madame la ministre, de compter sur la bonne volonté des dirigeants de l'audiovisuel public pour mener des coopérations « par le bas vieille expérience des contrats d'objectifs et de moyens (COM) nous a malheureusement instruits quant à la sincérité des engagements qui peuvent être pris par les uns et par les autres. Je me permets de partager avec vous, madame la ministre, le fruit de cette expérience la volonté de travailler ensemble exprimée par les dirigeants de l'audiovisuel public n'est jamais aussi aiguë que lorsque se profile le renouvellement de leur mandat ou la définition de la trajectoire budgétaire Hélas, en cette matière également, « les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent », comme aurait dit un grand acteur et connaisseur de notre vie démocratique. Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours des débats, mais les engagements pris dans les COM sont souvent peu suivis d'effets.

Il est inhabituel qu'une initiative parlementaire propose de modifier significativement la loi du 30 septembre 1986. C'est, je le crois, une chance pour le Gouvernement, qui ne saurait être accusé de poursuivre quelques desseins politiques. Sachez par ailleurs, madame la ministre, que nous sommes ouverts pour faire évoluer ce texte. Nous l'avons déjà fait concernant les modalités de nomination du président de France Médias. Nous pourrions le faire également concernant d'autres dispositions. Je pense, en particulier, à la vente des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions sportives ou au soutien au développement du DAB+,

il le sera d'autant moins si le Gouvernement n'entend pas intégrer la question du financement dans une vision plus globale, qui porterait également sur l'organisation et la gouvernance. Il y a aujourd'hui un chemin pour préserver notre souveraineté audiovisuelle, et nous souhaiterions l'emprunter ensemble, madame la ministre. Au moment où Mme la Première ministre appelle de ses voeux la recherche de majorités de projets, nous répondons favorablement à cet appel en vous tendant la main à notre tour. La parole est

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite de nouveau remercier le président de notre commission, Laurent Lafon, d'avoir pris l'initiative de déposer cette proposition de loi. C'est une proposition de loi sénatoriale, ce qui veut dire qu'elle est très équilibrée. Le caractère limité du temps imparti à la discussion des propositions de loi imposait de faire des choix, en ce qui concerne tant les sujets traités que le nombre de dispositions retenues. Comme nous l'a dit un acteur reconnu du monde des médias, le Sénat a montré qu'une réforme très ambitieuse pouvait être conduite au moyen d'un texte ne comportant qu'un nombre restreint d'articles. Le débat pour savoir si une réforme de la loi de 1986 est possible ou non est clos. Non seulement cette réforme est possible, mais elle est indispensable, et le plus tôt sera le mieux Si notre texte a reçu un si bon accueil de la part des grands acteurs français de l'audiovisuel, c'est aussi, madame la ministre, parce qu'il a pu bénéficier du travail réalisé par votre collègue Franck Riester voilà trois ans. Ce texte est donc aussi un peu le vôtre Pourquoi sommes-nous tant attachés à ce texte ? Parce qu'il permet d'abattre quelques mythes et de rappeler certaines réalités, sur lesquelles je souhaiterais maintenant revenir. Premier mythe, nous entendrons encore ce soir, je n'en doute pas, de la part de ceux qui ont fait si peu pour accompagner les transformations de l'audiovisuel public, que nous serions opposés au service public et que notre projet aurait pour objectif d'en réduire les moyens. La réalité est très différente, comme le démontre la proposition de loi. Nous sommes, au contraire, très attachés à l'existence d'un audiovisuel public fort, indépendant et s'adressant à tous les Français. S'il nous arrive de formuler des regrets, voire quelques critiques, c'est que nous considérons, comme le Président de la République en son temps, que l'audiovisuel public n'est pas exemplaire, ou tout du moins qu'il conserve des marges de progression pour développer des programmes plus originaux, pour veiller à l'impartialité de son information et pour s'astreindre à une gestion économe des deniers publics. Nous sommes également opposés, c'est un fait, à la politique du « quoi qu'il en coûte », y compris en matière d'audiovisuel public.

en allant plus loin sur les évolutions de structures et en renouvelant profondément son offre de programmes. L'objectif de cette proposition de loi est de permettre l'émergence de trois ou quatre grands groupes français des médias, qui pourront tenir leur rang en Europe. L'audiovisuel public doit faire partie de ces champions. Deuxième mythe, les mutualisations entre les sociétés de l'audiovisuel public donneraient satisfaction et il ne faudrait surtout rien changer. Ce deuxième mythe a peu de partisans parmi ceux qui connaissent la réalité des coopérations menées par les sociétés de l'audiovisuel public. Lors de son audition, le président de l'Arcom, Roch-Olivier Maistre, a ainsi déploré l'absence de coopérations éditoriales entre les équipes de France 3 et celles de France Bleu dans les matinales communes. Il a aussi regretté la persistance de programmes distincts pour la radio et la télévision s'agissant de France Info. J'ajouterai, pour ma part, qu'il est de plus en plus incompréhensible de maintenir autant de rédactions distinctes au sein de Radio France et de France Médias Monde. De même, on peine à comprendre pourquoi, à une exception près, les équipes de France 3 et de France Bleu en région n'ont toujours pas été regroupées dans des locaux communs. Les mutualisations ne peuvent continuer à avancer à ce rythme. Or, pour changer de tempo, rien de tel que de nommer un chef d'orchestre. J'en viens donc au troisième mythe : le regroupement de l'audiovisuel public serait inutile, coûteux et chronophage. Ce troisième mythe est évidemment le plus facile à démonter. L'éparpillement de l'audiovisuel français est un fait unique en Europe. Il montre chaque jour ses limites. Pourtant, certains n'ont de cesse de trouver cela formidable. Il est vrai que cette structuration n'a pas que des défauts, puisqu'elle permet la multiplication des présidences, des directeurs, des rédactions, des correspondants à l'étranger, des sites internet, des directions régionales et locales. Abondance de biens ne qui peut croire, à un moment où on leur demande autant d'efforts, que les Français vont accepter éternellement un tel laisser-aller ? Les appels à la privatisation se multiplient, il n'est plus possible de le nier. Pourtant, aucun compte n'est demandé à France Télévisions pour l'échec de Salto, qui a coûté au moins 80 millions d'euros, ni pour l'audience dérisoire de la chaîne France Info, qui coûte également des dizaines de millions d'euros chaque année. Nous reviendrons sur le prétendu coût de la holding. J'observe cependant que les partisans du surestiment ce coût, sans jamais le chiffrer, tandis qu'ils oublient toujours d'évoquer les économies considérables qu'elle permettrait de réaliser. Je terminerai en évoquant un quatrième mythe : les éditeurs de programmes français seraient très satisfaits de leur situation actuelle et ne demanderaient aucune réforme. Pour les avoir tous rencontrés de nombreuses fois au cours des derniers mois, je puis vous assurer qu'il n'en est rien. Qu'il s'agisse de la réglementation concernant la visibilité appropriée, les événements d'importance majeure, la production indépendante, la publicité ou le développement du DAB+, l'impatience a depuis longtemps cédé la place à l'exaspération, quand ce n'est pas à la colère pour les plus exposés à la concurrence des plateformes. Le Sénat ne peut se résigner à voir un secteur d'excellence français sombrer dans l'indifférence avec la complicité de tous ceux qui trouvent intérêt à s'allier avec les plateformes. Nous croyons, au contraire, à l'action publique et nous formons le voeu, madame la ministre, que l'élan réformateur porté par le Président de la République pourra également atteindre les rivages de l'audiovisuel français. La parole est à Mme

Monsieur le président, monsieur le président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication- cher Laurent Lafon -, monsieur le rapporteur- cher Jean-Raymond Hugonet -, mesdames, messieurs les sénateurs,

Cette proposition de loi témoigne, je le crois, de notre attachement commun à un audiovisuel public fort. Il est important de le rappeler à l'heure où certains remettent en cause son existence et plaident pour sa privatisation. Rappelons tout d'abord que, à l'issue de l'ambitieux plan de transformation mis en oeuvre ces dernières années, les résultats de l'audiovisuel public sont meilleurs que jamais. Celui-ci s'impose en effet comme le premier média des Français, en radio comme en télévision : 50 millions de téléspectateurs regardent les programmes de France Télévisions chaque semaine Radio France est écoutée chaque jour par plus de 15 millions d'auditeurs ; la part d'audience d'Arte a atteint un niveau historique ; chaque semaine, à travers le monde, Radio France internationale (RFI), France 24 et Monte-Carlo Doualiya rassemblent 260 millions de personnes.

En 2020, c'est vrai, le Gouvernement avait présenté un projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique. Avec ce texte, il entendait favoriser les coopérations entre France Télévisions, Radio France, France Médias Monde (FMM) et l'Institut national de l'audiovisuel (INA) au travers de la création d'une holding. La crise sanitaire a interrompu ce projet, mais pas l'accélération des coopérations. Cette démarche a porté ses fruits. Le média global France Info, qui est devenu le premier site d'information en ligne en France, est le fruit de la coopération entre toutes ces entreprises. Sa couverture quotidienne a doublé en cinq ans. En ce qui concerne la proximité, France Bleu et France 3 ont lancé une plateforme commune sous la marque « Ici » et ont groupé leurs forces. Depuis 2020, la plateforme Radio France rassemble toute l'offre de podcasts du service public. Elle est passée voilà un an devant Apple Podcasts. Un podcast sur deux qui est écouté aujourd'hui en France est un podcast de l'audiovisuel public. Les entreprises ont créé ensemble Culture Prime, offre culturelle commune sur les réseaux sociaux, et l'offre d'éducation Lumni. Il y a aussi des coopérations moins visibles, dites de gestion, mais qui n'en sont pas moins très importantes, par exemple la mise en place d'un club pour des achats groupés ou la coopération en matière de cybersécurité. Ces projets communs reposent sur une gouvernance souple et agile, qui permet aux équipes de définir ensemble les modalités les plus pertinentes de coopération, projet par projet. Cette agilité est un atout pour répondre aux nouveaux défis,

face à la multiplication des fausses nouvelles et des manipulations. Ce « chaos informationnel », pour reprendre les mots de Christophe Deloire, de Reporters sans frontières, s'est accéléré depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je pense aussi à la place prise par les plateformes, qui ont encore gagné du terrain depuis la crise sanitaire. Il y a donc urgence à accélérer également sur le numérique. Dès mon arrivée au ministère de la culture, en mai dernier, j'ai souhaité poursuivre et amplifier une dynamique qui porte ses fruits, en engageant rapidement les travaux de préparation des nouveaux contrats d'objectifs et de moyens. J'ai fait part de ma volonté de signer des contrats synchronisés entre eux et sur la durée de la mandature, à savoir cinq ans, de 2024 à 2028, au lieu de trois ans précédemment, afin de garantir aux sociétés la visibilité dont elles ont besoin pour faire face à ces défis.

J'ai relevé un large consensus sur cinq enjeux prioritaires : information, proximité, création, jeunesse et numérique. J'ai aussi pu constater l'engagement et la disponibilité totale des entreprises pour coopérer au service de ces priorités. L'approfondissement des coopérations sera donc un axe majeur des nouveaux contrats. Les parties prenantes que j'ai consultées ont formulé énormément de propositions très précises sur la détection des fausses informations, les investissements technologiques, la recherche et le développement, la mutualisation de la formation, etc. Pour la première fois, un contrat spécifique signé par toutes les entreprises sera consacré aux coopérations dans les COM, avec un calendrier de mise en oeuvre, des objectifs précis et des indicateurs. Des leviers pour renforcer le pilotage peuvent être identifiés. Un conseil stratégique des présidents de l'audiovisuel public pourrait se réunir mensuellement et se décliner avec des réunions des membres des comités exécutifs sur les sujets majeurs. La part variable de la rémunération des dirigeants pourrait par ailleurs davantage dépendre de leur capacité à mener à bien les chantiers de coopération. Voilà, concrètement, comment encourager les coopérations entre les entreprises au service d'une ambition forte pour lutter contre la désinformation, pour rapprocher les offres numériques, pour développer l'offre de proximité et pour toucher de nouveaux publics, notamment les jeunes. Les coopérations ne sont pas une fin en soi, et leur succès dépend avant tout de la clarté des objectifs. Un grand meccano institutionnel ne m'apparaît ni nécessaire ni prioritaire. Je suis convaincue qu'une véritable ambition pour l'audiovisuel public peut reposer sur des coopérations par projet et sur la confiance dans les dirigeants nommés par l'Arcom et dans leurs équipes, sans accroître les rigidités ni courir le risque de perdre en souplesse organisationnelle. Les travaux avancent très bien, et mon souhait est que ces contrats d'objectifs et de moyens 2024-2028 soient soumis pour avis au Parlement et au régulateur à l'automne prochain, pour les finaliser avant la fin de cette année.

en mobilisant l'énergie des entreprises sur des réorganisations de structure au détriment des priorités urgentes. Bref, c'est « une machine à perdre son temps », pour reprendre les mots de Pascal Rogard, directeur général de la Dans le rapport que vous avez publié en juin 2022, lequel préconisait une fusion, monsieur le rapporteur, vous indiquiez vous-même avoir « entendu les avis de nombreux experts auditionnés, qui s'interrogeaient sur l'intérêt de créer une holding compte tenu de la complexité de ce type de structure, qui ajoute une couche supplémentaire, avec le risque de multiplier le nombre des décideurs au lieu de le réduire. » Voilà qui est très clair ! Vous l'avez très bien dit vous-même, la création d'une holding induirait très certainement une complexification des processus et des coûts supplémentaires. J'ai moi aussi échangé avec de nombreux experts, et tous étaient plutôt sceptiques sur la holding, craignant que cette couche supplémentaire ne ralentisse finalement l'élan engagé en matière de coopération, qui s'approfondit et s'accélère. Monsieur le sénateur Hugonet, votre rapport évoquait la nécessité de « changer de cap », mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez changé de cap depuis Pour ma part, je ne serai pas favorable aux dispositions qui créent une société holding, car, si je partage l'ambition que vous nourrissez pour l'audiovisuel public, je ne partage pas le chemin que vous proposez pour servir cette ambition. La proposition de loi comporte un second volet relatif à la souveraineté audiovisuelle. C'est une priorité de notre action, et je veux rappeler ici quelques-unes des avancées majeures enregistrées depuis six ans dans ce domaine.

doivent financer la création française et européenne à hauteur de 20 % du chiffre d'affaires qu'elles réalisent en France. Leur investissement devrait représenter, chaque année, un surcroît de financement de l'ordre de 300 millions d'euros, qui viendra s'ajouter à la contribution, encore majoritaire et, bien sûr, déterminante, des chaînes historiques. Puisque c'est l'un des objectifs de ce texte, je rappelle que nous avons également donné plus de marges de manoeuvre aux chaînes traditionnelles : en les autorisant à faire de la publicité segmentée, ainsi que, à titre expérimental, de la publicité pour le cinéma ; en assouplissant l'encadrement de la diffusion de cinéma à la télévision en leur donnant les moyens de mieux rentabiliser leurs investissements dans la création. Vous le savez, monsieur le rapporteur, notre réforme des obligations de financement de la production audiovisuelle et cinématographique résulte d'un accord politique récent sur la définition de la production indépendante. est issu de la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique, dont vous étiez également rapporteur, monsieur Hugonet. De nombreux acteurs ont signé des accords en se fondant sur cet équilibre. Nous ne souhaitons pas le remettre en cause. Nous avons apporté des réponses à de nouveaux défis qui menacent la souveraineté audiovisuelle. Vous le savez, les grandes plateformes étrangères concluent des contrats avec les constructeurs d'équipements pour être mises en avant, que ce soit sur l'écran d'accueil des téléviseurs connectés ou sur la télécommande. Notre service public et nos acteurs nationaux, qui contribuent au pluralisme et à la diversité culturelle, sont de moins en moins visibles et accessibles dans ces nouveaux environnements. C'est pourquoi nous avons introduit des obligations de mise en avant des services audiovisuels d'intérêt général dans ces environnements. La mise en oeuvre de ces obligations par l'Arcom, notamment la définition des services d'intérêt général, est en cours, dans la concertation. Vous proposez de figer les choses dans ce texte. Je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure voie. Comment ne pas évoquer aussi rapidement la modernisation de la régulation et la création de l'Arcom, le renforcement de la lutte contre le piratage des oeuvres et programmes audiovisuels, la protection des catalogues cinématographiques et audiovisuels en cas de cession à un acteur étranger, ou encore le droit voisin des éditeurs de presse, combat que la France a porté avec beaucoup de force ? Enfin, j'ai annoncé récemment, à Cannes, l'identité des lauréats de l'appel à projets « La grande fabrique de l'image », dans le cadre du plan d'investissement France 2030. Cette initiative inédite, dotée de 350 millions d'euros, doit faire de la France un leader des tournages, de la production de films, séries et jeux vidéo, de la postproduction, des effets visuels et de la formation aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Il s'agit, là encore, de défendre pleinement notre souveraineté audiovisuelle et culturelle.

de la liste des événements d'importance majeure, pour garantir l'accès du plus grand nombre de téléspectateurs aux manifestations sportives, en particulier féminines. Je salue, sur ce sujet, l'engagement de David Assouline. Nous devons aller plus loin, et je partage pleinement avec vous l'objectif de soumettre les plateformes numériques aux mêmes obligations que les services de télévision.

Je partage aussi certaines propositions en faveur de la modernisation de la télévision numérique terrestre (TNT). La diffusion hertzienne demeure le seul mode de diffusion gratuit, souverain et anonyme, et les chaînes de la TNT portent encore l'essentiel du financement de la création. C'est pourquoi je soutiens les dispositions adoptées en commission, l'initiative de Mme Morin-Desailly, sur l'ultra-haute définition. J'ai moi-même récemment saisi l'Arcom pour permettre à France Télévisions d'offrir à nos concitoyens une diffusion des jeux Olympiques de 2024 en ultra-haute définition. Je soutiens aussi, en matière de radio, le déploiement du DAB+, cette norme de diffusion souveraine plus économe en ressources. Le texte qui vous est soumis nous paraît soulever quelques difficultés juridiques, mais le sénateur Julien Bargeton a proposé une rédaction de substitution qui permettrait de les surmonter. Nous aurons l'occasion de reparler de ces articles, ainsi que de ceux que je n'ai pas mentionnés. Je veux conclure en vous remerciant toutes et tous, mesdames, messieurs les sénateurs, de votre mobilisation constante- pour certains d'entre vous, depuis de nombreuses années -sur ces enjeux : vos travaux, votre expertise et votre engagement

jamais notre société n'a eu autant besoin de repères clairs et innovants dans la diffusion d'informations, de culture et de divertissement. L'audiovisuel public a cette lourde tâche de fournir une information indépendante, indispensable à la vie démocratique, ainsi que des divertissements qui doivent permettre la diffusion de contenus culturels, sportifs et éducatifs vers une population qui en serait éloignée. Il doit prolonger l'enseignement public dans l'élévation des individus au rang de citoyens éclairés. Depuis la loi Léotard de 1986, s'il y a eu quelques évolutions, il n'y a pas eu de grande réforme qui aurait permis à l'audiovisuel public de mieux répondre à la révolution numérique et aux offensives des grands groupes privés étrangers, qui ont su bien mieux exploiter les nouvelles technologies numériques.

Aussi cette proposition de loi de Laurent Lafon propose-t-elle une réforme attendue et nécessaire de l'audiovisuel public et de sa souveraineté. Elle soulève les inquiétudes et les oppositions de tous les conservatismes du secteur, qui devrait, au contraire, avoir l'ambition de s'adapter au contexte d'avancées technologiques et de concurrence qu'imposent les nouveaux modes de « consommation culturelle », comme on les appelle, et de recherche d'intégrité des informations. L'ambition du texte est grande. Il s'agit de retrouver une stratégie et une capacité d'innovation depuis longtemps perdues. En rassemblant les quatre entreprises nationales de l'audiovisuel public dans une même structure, nous obligerons les différentes grammaires à se rencontrer et à apprendre à faire sens commun. Sensibles à un développement structurel de l'audiovisuel public, les auteurs de la présente proposition de loi entendent supprimer les contrats d'objectifs et de moyens pour créer des conventions pluriannuelles stratégiques. En assumant le choix de détenir la totalité du capital de ce groupement, l'État réaffirme son engagement pour la pérennité et son souci de sécurité pour nos médias publics. Il est certain qu'une telle proposition bousculera les habitudes et les méthodes de travail. L'enjeu est alors de respecter la subsidiarité et de faire confiance. La diversité de la composition du conseil d'administration permet d'y veiller. Enfin, faire oeuvre pour l'audiovisuel ne peut se faire sans un travail collaboratif avec le secteur privé. En demandant aux chaînes payantes de laisser une place à l'audiovisuel public, notamment lors des événements sportifs, cette proposition fait place au commun et amorce la fin de l'égoïsme concurrentiel. Pour ma part, si j'ai applaudi à la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, qui était injuste et insuffisante,

Parce que cette proposition de loi reconnaît, dans l'audiovisuel public, un vecteur de connaissances, de créativité, de critiques, de divertissements et d'enseignements, le groupe RDSE ne se prononcera qu'à l'issue des débats sur ce texte que, pour ma part, je soutiens.

En réalité, je pense que la détermination élyséenne à faire une réforme de l'audiovisuel public avait disparu en 2019.

trente-sept ans, on aménage à la marge, mais on n'a pas voulu regarder les choses en face. Or le paysage a changé, en Europe, dans le monde, avec les plateformes, avec la concurrence du privé. Tout a changé

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». Cette initiative non concertée de notre collègue Laurent Lafon en est, malheureusement, une nouvelle illustration. Le 31 mai dernier, à la suite de l'adoption d'une loi pour la préservation du journalisme par l'assemblée de Californie, le directeur de la communication politique de Facebook-Meta a menacé de supprimer le fil d'actualité de Facebook, « plutôt que de payer pour une caisse noire », comme il l'a écrit Depuis une dizaine d'années, nous sommes devenus les spectateurs de la transformation du paysage médiatique international, avec l'essor des plateformes de service de vidéo à la demande, le développement des réseaux sociaux et la croissance du marché publicitaire comme source de financement, notamment des compétitions sportives. Il en résulte une très forte concentration médiatique, dominée par quelques géants dont les règles internes ont presque force de loi. En 2025, le marché mondial de la publicité pourrait franchir le cap de 1 000 milliards de dollars, soit le PIB des Pays-Bas. Les trois sociétés Google, Facebook et Amazon détiennent désormais plus de 50 % de ce marché. Cette position ultradominante leur permet d'exercer un chantage sur les parlements à travers le monde. En France, la commission d'enquête sénatoriale conduite par notre collègue David Assouline a mis en lumière la concentration médiatique également à l'oeuvre dans notre pays, ainsi que ses conséquences sur la liberté de la presse. Certes, on n'y découpe pas les journalistes à la tronçonneuse, comme en Arabie Saoudite, pas plus qu'on ne les détient arbitrairement pour motif d'espionnage, comme en Russie, mais on les licencie, on les démet de leurs fonctions. alimente la défiance populaire à l'encontre de ceux qui nous informent : 62 % des Français ne feraient pas confiance aux journalistes et 41 % d'entre eux s'informeraient dorénavant prioritairement les réseaux sociaux, sociaux, où les contenus journalistiques côtoient les commentaires dépourvus de fondements factuels, noyés dans une masse d'informations anecdotiques et personnelles. Dans ce contexte, notre collègue Laurent Lafon nous propose une « stratégie ambitieuse et globale », rédigée sur sa seule initiative. En fait de stratégie et d'urgence, ce texte propose de renforcer les positions dominantes, à l'opposé des recommandations de la commission d'enquête que j'ai citée, pour offrir une nouvelle fenêtre de fusion entre TF1 et M6 et pour adapter les règles de droits de diffusion des événements sportifs majeurs, qui favorisent Canal+. Pis, après la suppression de la redevance l'été dernier, la création d'une holding réunissant quatre acteurs de l'audiovisuel public constitue l'autre pilier de cette stratégie. Cet étage supplémentaire nous promet des années d'immobilisme, à l'heure où l'évolution du secteur nécessite de la souplesse, de l'adaptation et de la rapidité décisionnelle. Cela va évidemment affecter les moyens destinés à la réalisation de missions de service public. Les auteurs-réalisateurs et les cinéastes Aujourd'hui encore, France Télévisions est le deuxième diffuseur de films après Canal+, et près de 40 % des droits perçus par les auteurs proviennent de sociétés publiques ... À quoi bon renforcer notre souveraineté audiovisuelle si cela fragilise l'exception culturelle française ? ne parle pas du mode de désignation du président de la holding par décret présidentiel, absolument contraire au projet de directive sur la liberté des médias présenté par la Commission européenne en septembre 2022 Nous y sommes fortement opposés. L'information n'est pas un bien comme les autres. Les entreprises de médias devraient être soumises non pas au droit de la concurrence, mais à des règles spécifiques, destinées à garantir le pluralisme et l'indépendance des rédactions. L'urgence, bien sûr, c'est de réviser la loi de 1986, qui est devenue obsolète. L'urgence, ce n'est pas d'ajouter une strate supplémentaire, non budgétisée, qui « ne coûterait rien », selon notre rapporteur, mais qui viendrait, de fait, amputer le financement de l'audiovisuel public. L'urgence, ce serait d'allonger les contrats d'objectifs et de moyens et de renforcer les synergies, mais ce serait aussi et surtout de garantir des mesures pérennes pour l'audiovisuel public. La Lolf doit prévoir un financement, comme le recommandent également les auteurs du rapport d'information publié le 7 juin dernier par l'Assemblée nationale. Du côté de la publicité, des gisements fiscaux existent pour financer l'audiovisuel public. La Californie nous en montre le chemin. L'urgence est au renforcement des moyens d'informer, non à la restriction budgétaire.

En février 2023, Delphine Ernotte et Sibyle Veil se sont prononcées pour un document stratégique unique de l'audiovisuel. Depuis lors, les coopérations

un outil équivalent à la holding. En effet, partager une ambition similaire n'empêche pas de réfléchir à des outils différents

accroissant sans cesse leur domination financière, qui les fait rivaliser avec les États les plus puissants du monde, au point de s'émanciper des règles et du droit, la droite sénatoriale a décidé de légiférer sur le service public de l'audiovisuel- en l'affaiblissant.

l'édition,, () et Europe 1, restructurés pour servir une ligne idéologique trumpiste à la française -, vous, la droite sénatoriale, avez décidé de montrer du doigt le service public de l'audiovisuel

alors même que le financement de l'audiovisuel public n'est plus assuré sur le moyen et le long terme du fait de la suppression de la redevance. Vous autorisez la troisième coupure publicitaire des fictions après vingt heures, satisfaire le privé. Vous ramenez à deux ans le délai de revente d'une fréquence après son acquisition, alors que c'est le Sénat, sur ma proposition, soutenue par Catherine Morin-Desailly, qui l'avait porté à cinq ans pour éviter les reventes spéculatives. Vous attaquez de nouveau la diversité de la production indépendante. Vous ouvrez le label Sieg (services d'intérêt économique général) aux sociétés privées pour une visibilité égale à celle des sociétés publiques, alors qu'elles ne remplissent aucune mission de service public.

équivalents temps plein (ETP) à Radio France ces dernières années et des baisses budgétaires régulièrement imposées par les gouvernements du président Macron, soit 193 millions d'euros pour la période 2018-2022. Vous proposez donc- quelle nouveauté, quelle innovation, quelle audace ! -de créer ... une holding. Et vous osez dire que c'est pour mieux faire face aux plateformes étrangères et à la concurrence. J'imagine déjà la frayeur au sein des d'Amazon, de Netflix, d'Apple ou de Google Ils doivent encore être en cellule de crise pour élaborer la riposte, la peur au ventre ... J'imagine le vent de panique des propriétaires des fournisseurs d'accès du numérique- Patrick Drahi chez SFR, Martin Bouygues et Xavier Niel soit dit en passant, sont aussi fournisseurs d'accès au service public -, qui détiennent une part grandissante des médias privés français et contrôlent de façon verticale toute la chaîne de production de la valeur ! J'imagine même l'effroi de M. Bolloré, demandant conseil à son confesseur qui, paraît-il, ne le quitte plus ! Je les imagine tous tourner en rond, en se

bureaucratique, une structure de plus coûtant des dizaines de millions d'euros de dépenses supplémentaires pour payer des super-chefs qui dirigeront des chefs, lesquels dirigent eux-mêmes d'ores et déjà des sous-chefs. désorganiserait ce qui a mis du temps à se stabiliser. Elle concentrerait l'énergie de ces sociétés sur une réorganisation administrative interne, au moment où ladite énergie devrait être tout entière dirigée vers l'action, consolider l'offre créative dans les domaines de la fiction comme du documentaire, de l'information et du sport, qui sont les valeurs ajoutées de l'offre en continu et en direct, pour investir dans la révolution numérique, s'y former et se préparer à ses prochains bouleversements induits par l'intelligence artificielle

progressive sur l'impôt sur le revenu, directement affectée, comme mon groupe l'avait proposé. Il faut en effet lui donner les moyens de résister à la concurrence des Gafam et des grands groupes privés qui détiennent les médias dans notre pays, en légiférant et en décidant de règles et de régulations nouvelles,

dans le cimetière de l'audiovisuel français ! Il y va de la démocratie. Avec mes camarades du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, je lance un appel urgent à cette prise de conscience. Une grande illusion produit ses effets, car il y a un paradoxe : la multitude des offres, des titres et des chaînes numériques cache la réalité de la concentration de la propriété au profit d'un nombre réduit

de le souligner, à l'heure où ce service public est attaqué de toutes parts. L'enjeu des inégalités sociales liées à la multiplicité des services payants par abonnement, celui de la concentration des médias ou encore de la désinformation croissante rendent d'autant plus essentiel et urgent

est le signe d'une démocratie qui fonctionne, d'un accès à la culture et au savoir pour tous et toutes. C'est à ce titre que nous accueillons positivement la proposition concernant les droits

-, ce texte risque de ne susciter qu'une nouvelle inertie des institutions publiques. Par ailleurs, les coopérations entre les différentes entreprises de l'audiovisuel, que ce projet de holding

sera le mieux à même de garantir l'indépendance des organismes de l'audiovisuel et la prévisibilité de leurs ressources. En revanche, rien dans l'exposé des motifs ne permet de savoir quelle serait la nature de cette mesure. S'il s'agit de pérenniser l'attribution d'une fraction

taxe affectée : son montant étant fixé en loi de programmation des finances publiques, elle ne permet en aucun cas de garantir le respect des engagements pluriannuels de l'État. En outre, la TVA constitue la mesure fiscale la plus anti-redistributive, fait peser l'effort sur la propension de consommation plutôt que sur l'épargne, désavantageant, de fait, les foyers les plus modestes. Pourtant, le retour d'une contribution à l'audiovisuel public, payée par tous les Français en fonction de leurs revenus, serait totalement justifié pour maintenir un lien fort avec les citoyens et garantir

Nous déplorons ce choix réalisé en faveur des chaînes privées, qui cherchent toujours à obtenir une plus grosse part du gâteau publicitaire. Sans compensation financière garantie, une telle disposition fragiliserait encore davantage l'audiovisuel public. À nos yeux,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, pourquoi mettons-nous autant de temps dans notre pays pour réaliser les réformes structurelles nécessaires et nous adapter à un monde en perpétuelle évolution ? Je pense ainsi au temps qu'il aura fallu pour imposer un cadre régulant et sécurisant l'espace numérique.

les changements et risques systémiques induits par les nouvelles technologies et l'accélération des innovations lors des quinze dernières années auraient dû inciter les gouvernements successifs à réagir rapidement et, à défaut, à écouter davantage le Parlement, en particulier les propositions du Sénat sur l'audiovisuel. Ce n'est pas comme si rien n'avait été fait ! Notre commission de la culture et ses rapporteurs successifs, dont j'ai eu l'honneur de faire partie, ont demandé sans relâche la réforme de la redevance qui s'imposait- les pays voisins l'avaient réalisée ! -, ainsi que l'indispensable évolution du cadre législatif et réglementaire, conçu pour un monde hertzien en voie de disparition.

pour adapter notre audiovisuel à l'heure du tout-digital. On le sait, il y a belle lurette que la loi de 1986 est obsolète et que nos règles de concurrence sont dépassées. Le récent échec de la fusion entre TF1 et M6 en est la dernière et consternante illustration. Face à la toute-puissance des Gafam, pour assurer notre modèle de création un pôle audiovisuel privé fort, tout comme un pôle audiovisuel public fort. Sur ce point, j'ai toujours dit que la réforme de 2009 était restée au milieu du gué.

qui se concentre sur les questions de gouvernance : la création d'une holding regroupant France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Cet outil important, nous le voulons souple- nous n'étions pas favorables à la fusion, pensant qu'elle cannibaliserait les énergies et ferait perdre du temps. Il permettra de permettra de regrouper les forces et les énergies de l'audiovisuel public, avec des équipes engagées dans des coopérations encore plus nombreuses, pour réaliser ensemble les investissements nécessaires. Ces investissements serviront à aller chercher les publics, notamment les jeunes, face à la concurrence, à développer des outils tels qu'une grande plateforme de l'audiovisuel public- je l'ai régulièrement évoquée en tant que membre du conseil d'administration de France Télévisions. J'ai toujours alerté, d'ailleurs, sur l'échec annoncé de Salto. L'idée de départ de Delphine Ernotte était bonne, mais, face aux géants, cette plateforme regroupant des financeurs publics et privés de la création ne pouvait se réduire à trois acteurs.

L'autre volet de la proposition de loi vise à réduire les asymétries qui pénalisent les médias historiques. Je n'ai pas le temps de développer ce sujet, mais je me réjouis notamment du rétablissement de l'équité en matière de règles de diffusion des événements sportifs majeurs.

qui a encore quelques années devant elle, je suis sensible aux avancées que comporte le texte à cet égard. Je remercie aussi le rapporteur d'avoir prévu un article 14 qui impose progressivement la compatibilité des nouveaux téléviseurs avec l'ultra-haute définition Cette disposition, que j'avais fait adopter en 2021, avait malheureusement été censurée de manière incompréhensible par le Conseil constitutionnel, pour des raisons de procédure. Je regrette, en revanche, que mes amendements relatifs à l'accès des chaînes de télévision

qui fixe le principe d'une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante et prévisible pour l'audiovisuel public. Encore faut-il que cela se traduise dans les faits en loi de finances, ainsi qu'au travers d'une loi organique. En l'absence de certitudes, je suis assez réservée sur le plafonnement de la publicité ; pourtant, je rêve d'un modèle totalement libéré. Le problème

heures. On comprendra donc que, pour le moment, le financement de l'audiovisuel demeure aléatoire et périlleux. Cette question est loin d'être anecdotique à l'heure où le projet de règlement européen relatif à la liberté des médias est en débat.

Il serait tout de même paradoxal que la France ne montre pas l'exemple en assurant à son audiovisuel la ressource permettant sa pérennité et, surtout, son indépendance. Car il y a une vraie différence entre une dotation publique et une dotation d'État, entre une ressource affectée et une ligne budgétaire calibrée selon le bon vouloir de Bercy ! Cette différence, nos partenaires allemands d'Arte n'ont pas manqué de la souligner lorsque nous avons supprimé la redevance. Pour eux et pour nombre d'observateurs

Je vous remercie, Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis trente ans, le paysage audiovisuel français ne cesse de se transformer. Notre pays est caractérisé par une grande diversité et une longue tradition de production cinématographique et télévisuelle. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Néanmoins, les nouveaux usages apparus tendent à privilégier les vidéos en ligne plutôt que les chaînes traditionnelles. Nous accordons tous une grande importance à notre service public audiovisuel. Des chaînes de télévision publiques, telles que France Télévisions et Arte France, fournissent un service de qualité, pluraliste et accessible à tous les citoyens. Elles ont un rôle clé dans la promotion de la culture, de l'éducation, de l'information et de la diversité. Cependant, l'évolution des habitudes de consommation des médias a eu un impact sur l'audiovisuel en France et a entraîné une baisse de la durée d'écoute des chaînes de télévision traditionnelles. Ensuite, avec l'essor de la concurrence internationale des plateformes de en ligne, comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, les téléspectateurs français ont désormais accès à un large éventail de contenus étrangers. Ces plateformes ont rassemblé 9,4 millions d'utilisateurs quotidiens en 2022. Cela crée une concurrence et un défi pour l'industrie audiovisuelle française, qui doit rivaliser pour attirer et fidéliser son public. Face à ces évolutions, la puissance publique est demeurée jusqu'à présent en retrait, peinant à réformer un cadre législatif posé en 1986 pour réguler un univers strictement national à une époque où internet n'existait pas. Il est clair que nous devons renforcer l'audiovisuel public et notre souveraineté audiovisuelle par une stratégie ambitieuse et globale. Pour cela, deux piliers ont été ciblés le regroupement de l'audiovisuel public, respectant l'identité de ses différentes composantes, et une révision significative de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Tel est l'objectif de la proposition de loi de notre collègue Laurent Lafon ; un objectif que nous partageons amplement. Je souhaite remercier également le rapporteur, Jean-Raymond Hugonet, de l'ensemble du travail réalisé. Mes chers collègues, en regroupant France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'INA au travers de la création d'une société holding, France Médias, nous assurons leur compétitivité et leur développement stratégique au niveau européen et international, tout en veillant à la cohérence et à la complémentarité de leurs offres de programmes.

Ce texte a un objectif clair : renforcer la qualité de la mission de service public de l'audiovisuel français, ainsi que sa souveraineté. Dans le contexte géopolitique actuel, l'enjeu est de garantir à nos concitoyens une information de qualité, tout en luttant contre les, ce qui est un véritable enjeu. Mutualiser les forces de ces entreprises sera donc synonyme de richesse médiatique et culturelle, mais aussi source de gains économiques. Il paraît cohérent de vouloir rassembler des entreprises qui, au nom de leur mission de service public, partagent les mêmes ambitions et ont des projets industriels similaires. Toutefois, cette mutualisation n'est pas synonyme de concurrence interne ; elle a bien pour objectif de mutualiser les logistiques et les investissements, afin de garantir un contenu gratuit et qualitatif. Ce point est fondamental. Prenons l'exemple de l'INA. Cette grande institution est freinée dans ses relations avec les autres entreprises à cause de son statut juridique. Au sein de la holding France Médias, elle gagnera en flexibilité et en efficacité. De plus, elle pourra prendre en charge la conservation des archives audiovisuelles diffusées de manière délinéarisée par les autres sociétés et les futures filiales de la holding. Pour ce qui concerne France Médias Monde, dont les journalistes et le réseau de correspondants offrent, en vingt et une langues, une information essentielle d'ouverture sur le monde et sur la diversité des cultures et des points de vue- je souhaite le souligner dans le contexte géopolitique actuel -, l'adoption de la proposition de loi permettra d'augmenter les synergies avec les autres chaînes publiques et, ainsi, d'accroître ses compétences à l'international. Cette proposition de loi permet également de reconnaître l'importance de l'innovation et des nouvelles technologies dans le paysage audiovisuel. Elle encourage la coopération entre les acteurs publics et privés, pour favoriser l'émergence de nouveaux formats et de nouvelles expériences pour les téléspectateurs. Elle permet à l'audiovisuel public de rester pertinent et attractif dans un environnement médiatique en constante évolution. Enfin, elle a le mérite d'aborder la question cruciale du financement, surtout après la suppression de la redevance public (CAP), nous garantissons un financement pérenne et équitable, sans faire peser une charge excessive sur les contribuables. Il est essentiel que chaque euro investi dans nos médias publics serve réellement à la promotion de notre culture, de notre histoire et de nos valeurs. En outre, ce texte garantit que les ressources nécessaires seront disponibles pour soutenir la production de contenus de qualité, la modernisation des infrastructures et le développement de nouveaux formats. En donnant davantage d'autonomie financière à nos médias publics, il garantit donc une information objective et équilibrée. de loi ne s'arrête pas à la création d'une holding. Elle prévoit aussi d'encadrer la concurrence étrangère, qui, du fait d'un manquement législatif, ne prenait pas en compte les évolutions concurrentielles audiovisuelles et numériques.

Les asymétries entre les chaînes et les plateformes numériques seront drastiquement réduites. C'est un point capital. L'industrie audiovisuelle française ne sera plus injustement pénalisée et pourra pleinement investir les marchés émergents. Pour conclure, mes chers collègues, cette proposition de réaffirmer notre attachement à la souveraineté audiovisuelle française ; de renforcer la mission de l'audiovisuel public français face à la désinformation et au contexte géopolitique mondial perturbé ; enfin, de définir une véritable vision pour l'audiovisuel public à partir d'orientations stratégiques claires, tout en veillant à la cohérence et à la complémentarité des offres

De nouveaux concurrents sont apparus : les grandes plateformes ont complètement changé les règles du jeu. De nouveaux modèles de consommation se sont développés ; les tablettes sont arrivées,

La télévision et la radio font partie de la vie quotidienne des Françaises et des Français. Elles participent à créer un socle commun- j'ose le mot -et sont un puissant vecteur culturel. Délivrer une information de qualité coûte cher, peut être copié instantanément et ne s'accompagne pas de droits d'auteur rémunérés. La souveraineté audiovisuelle doit permettre aux médias nationaux de délivrer une information de qualité, vérifiée, fiable et objective.

Franck Riester s'en était inspiré par la suite. Malheureusement, le projet de loi annoncé a fait les frais de la crise de la covid-19. La création d'une société de tête proposée par ce texte va dans le bon sens. Il s'agit de regrouper les forces de l'audiovisuel public une entité visible, cohérente et identifiée, qui regroupera France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'INA. Cette structure doit être la plus souple, la plus complémentaire, la plus réactive et la plus mutualisée possible

Évidemment, ce n'est pas au politique de décider de la grille des programmes, mais c'est au législateur de poser un cadre pour garantir la qualité de l'information, la diversité et la créativité culturelle, ainsi que pour permettre la diffusion des grands événements sportifs. L'audiovisuel public doit représenter toutes les sensibilités et toutes les opinions- Chaque Français doit pouvoir s'y reconnaître. Dans ce texte, si la question de la publicité est abordée, nous n'en sommes qu'au début d'un long débat. Comme beaucoup, je comprends l'argument consistant à expliquer que l'audiovisuel public ne peut fonctionner selon le même modèle économique que les chaînes privées, avec les mêmes enjeux et les mêmes priorités.

Les producteurs indépendants français comptent parmi les tout meilleurs au monde. Veillons à ne pas remettre en cause leur dynamisme et leur développement en touchant à la relation entre diffuseurs et éditeurs. et Territoires sont très attachés au maintien et au renforcement des émissions locales et régionales. Celles-ci représentent autant de relais d'information qui font le quotidien des territoires et de leurs habitants. Les journalistes doivent continuer à décrypter les actualités de terrain. De la même manière, notre audiovisuel public doit être le relais des territoires d'outre-mer. L'audiovisuel public doit être un repère, un modèle et un exemple. Il doit continuer d'être une ouverture sur le monde, sur la culture et sur la société. Notre rôle est de garantir sa singularité sur le long terme en proposant un cadre juridique stable et pérenne, qui permette de réduire les asymétries pénalisant nos acteurs de l'audiovisuel, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Ce texte est un bon signal. Il démontre notre attachement et notre préoccupation concernant l'audiovisuel français.